La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Chacun

Monsieur le Premier ministre, nos forces armées viennent de subir la perte tragique de treize militaires d'élite, en action de combat, au Mali. Nous nous inclinons devant leur sacrifice et nous rendons hommage à leur courage, celui de tous les hommes et femmes engagés sous les armes. L'opération dans laquelle nos soldats sont engagés a été autorisée par le Parlement, conformément à la Constitution, et nos commissions en sont tenues informées. Elle est légitime, a été décidée en plein accord avec les autorités du pays, et elle apporte un appui décisif à la force des Nations unies chargée d'oeuvrer à la stabilisation du Mali.

il est important que vous redisiez, aujourd'hui, devant le Sénat, les actions déjà menées par nos forces contre nos ennemis, dans le Sahel, le concours que nous apportent les nations partenaires et la coopération développée avec le Mali et ses voisins, pour construire la paix dans cette région, qui importe tant à notre sécurité.

m'associer au message de respect et de tristesse que vous venez de formuler, à l'intention de nos compatriotes qui servent sous les drapeaux, drapeaux, de leurs familles, de leurs compagnons d'armes, et à l'intention de tous ceux qui mesurent, parce qu'ils les connaissent et qu'ils en sont proches, le sacrifice que nos soldats sont susceptibles de faire, et l'engagement- l'engagement de toute une vie -qu'ils prennent en servant les armées françaises. Je le dis, monsieur le sénateur, à quelqu'un qui le sait mieux que d'autres, compte tenu des fonctions que vous avez exercées : nous pouvons être fiers de nos forces armées. Je le dis au Sénat, avec un profond respect et une immense admiration, alors alors que nous savons tous que les treize morts que nous devons déplorer dans cette opération de combat au Mali touchent particulièrement cette maison, cet hémicycle, en la personne de votre collègue, de notre ami, Jean-Marie Bockel. La France se bat au Mali. Plus exactement- j'ai souvent l'occasion de le souligner -, dire : « la France se bat au Mali », c'est dire, en vérité : « des hommes et des femmes se battent au Mali pour la France, pour y défendre sa sécurité, pour garantir la stabilité d'États amis, alliés et partenaires ». Elle se bat au Mali depuis que le précédent Président de la République a considéré qu'il était de l'intérêt de la France d'aller stopper cette avancée vers Bamako, qui menaçait de déstabiliser une région et de permettre la constitution d'une zone de non-droit, dans laquelle, nous le savons, des groupes armés terroristes se seraient organisés afin de pouvoir, ensuite, déstabiliser, non seulement la région, mais encore notre pays, y compris par des actions terroristes.

présente- par la force, par la capacité numérique de son engagement, par la compétence des forces armées qu'elle déploie sur ce territoire -, mais elle n'est pas seule.

participent-ils assez ? C'est une question délicate et nous avons, à l'évidence, un travail de conviction à mener avec nos partenaires européens- et, au-delà, avec nos alliés -sur l'intérêt commun que nous avons à faire prévaloir des zones de paix et de développement dans la bande du Sahel, sous peine d'avoir à subir chez nous, en Europe, et partout dans le monde, la déstabilisation que j'évoquais précédemment. Nous devons- c'est l'objectif fixé aux forces armées françaises qui participent aux opérations -, déstabiliser les groupes armés terroristes. Nous devons déstabiliser leurs caches d'armes, leurs routes d'approvisionnement. Nous devons réduire leurs points forts. Nous devons accompagner les armées des États concernés, notamment ceux du G5 Sahel, dans leur montée en puissance, indispensable pour garantir la paix. Nous devons aussi- nous le savons parfaitement, et ce n'est pas facile -faire en sorte que le combat ne soit pas simplement militaire, car, si le combat militaire est nécessaire, il n'est pas suffisant pour régler des questions qui se posent, parfois depuis très longtemps, dans cette région. Il y a donc tout un travail de stabilisation politique, qui revient souvent aux États concernés, et de développement économique et de perspective pour l'ensemble des populations. Ce que je veux dire, monsieur le sénateur, en vous répondant ainsi, c'est que le combat que nous livrons est un combat militaire dur

les risques auxquels s'exposent nos soldats, on ne les voit pas très bien, on ne les mesure pas complètement. Tous ceux qui s'engagent sous les drapeaux les connaissent ; cela ne rend pas le risque moins intense ni le chagrin moins fort, mais c'est un risque qui est connu et que prennent consciemment les jeunes gens qui sont au service de la France. Nous devons en être fiers et les célébrer ; nous devons accompagner ceux qui restent- les conjoints, les enfants, les parents -, les accompagner de la chaleur de notre fraternité ; et nous devons savoir que ce qui se joue là-bas est important pour nous ici, et que ce combat sera long et difficile. L'honneur d'une démocratie, c'est de faire en sorte que le pouvoir politique choisisse d'engager des troupes sur un théâtre d'opérations étranger lorsqu'il considère que c'est nécessaire ; c'est une lourde responsabilité et elle a été lourde pour tous ceux qui ont exercé ces choix. L'honneur d'une démocratie, c'est aussi de dire la fierté que représentent, pour nous tous, ces hommes et ces femmes. J'ai bien conscience, monsieur le président, qu'en disant ces mots je suis un peu maladroit, mais je veux vous dire, mesdames, messieurs les

dans la collision de deux hélicoptères au cours d'une opération de combat au Mali. Au nom de tous les collègues de mon groupe, je souhaite rendre hommage au courage de ces héros, qui ont péri ensemble au cours cette tragédie. Je tiens à honorer leur mémoire, et je veux adresser notre soutien le plus profond aux familles endeuillées. J'ai naturellement une pensée particulière pour notre collègue Jean-Marie Bockel et sa famille. À cet instant, alors qu'un hommage national sera rendu aux Invalides lundi prochain, il me paraît crucial de réaffirmer notre soutien aux 4 500 soldats engagés sur le terrain pour combattre le terrorisme islamiste qui nous frappe ici aussi, en France et en Europe. Par-delà les débats que certains voudraient engager sur la stratégie de la France dans la région du Sahel, je veux rappeler deux choses, simples et pourtant fondamentales : sans l'opération Barkhane, le Mali, pays ami de la France, serait aujourd'hui sous la domination de nos ennemis au Mali, la France fait face, trop seule, à l'organisation de l'État islamique dans le Grand Sahara. C'est d'ailleurs sur ce point que je souhaite vous interroger, monsieur le Premier ministre. Dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans la région du Sahel, alors que la France protège toute l'Europe au travers de cette opération, quelles initiatives comptez-vous prendre pour obtenir un soutien militaire renforcé de la part de nos alliés européens, qui sont, de fait, directement concernés ? Quelles initiatives diplomatiques et politiques, la France prend-elle auprès de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations unies,

dans les moments difficiles, mais aussi tout au long de l'année. Monsieur le sénateur, la France reste, plus que jamais, engagée aux côtés du Mali. À court terme, nos axes d'effort consistent d'abord à soutenir les armées locales et la force du G5 Sahel

La France veut mobiliser les Européens pour lancer la force Takouba, un déploiement de forces spéciales européennes, en accompagnement des Maliens. dit, M. le Premier ministre vient de le dire, la solution n'est pas que militaire, l'accord de paix doit être mis en oeuvre et nous devons progresser en matière de gouvernance et de développement. C'est au gouvernement malien qu'il appartient de jouer un rôle moteur son engagement à désarmer toutes les milices et à aller au bout du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion doit être suivi d'effets. La France est prête à aider les Maliens à faire face à la crise survenue le Premier ministre malien s'est rendu dans cette région et a permis la signature d'accords locaux, ce qui est un pas supplémentaire. Le retour de la sécurité et de la justice est impératif, mais il faut également traiter les causes profondes de la crise,

et solidaire, le Var vient de subir de nouvelles inondations dramatiques : nous déplorons cinq morts et des dégâts dont le montant devrait se situer entre 180 millions et 300 millions d'euros. À l'origine, comme c'est classiquement le cas dans le Var et dans tout le sud de la France, de violents orages de type cévenol, avec le ruissellement torrentiel qui en résulte. Pourtant, par l'un de ces mystères bureaucratiques dont notre pays fait ses délices,

Madame la ministre, combien de catastrophes vous faudra-t-il encore pour admettre l'urgence qu'il y a à lever les obstacles au déploiement d'une politique pérenne de prévention de l'inondation dans le sud du pays ?

décès, le bilan est lourd, et j'ai bien évidemment une pensée pour les proches des victimes. Je veux aussi saluer l'exceptionnelle mobilisation des forces de secours, des services de l'État, des opérateurs et des élus locaux, qui ont fait face, ce qui a permis que le bilan ne soit pas plus lourd. Bien entendu, le Gouvernement assurera un suivi attentif de l'ensemble des conséquences de ces intempéries. Le cumul des précipitations a été très important, ce qui a justifié le placement, par Météo France, de deux départements- le Var et les Alpes-Maritimes -en vigilance rouge. De fait, notre pays doit se préparer à vivre ce type de phénomènes de plus en plus souvent et de plus en plus intensément. C'est pourquoi il faut effectivement agir pour la prévention des inondations, et c'est ce que nous faisons, en particulier avec les programmes d'action pour la prévention des inondations, financés notamment par le Fonds Barnier. J'attends, pour les prochains jours, un rapport d'inspection de mon ministère, qui doit dégager des pistes pour mettre en oeuvre plus rapidement ces programmes d'action pour la prévention des inondations. Toutes les propositions seront bien sûr examinées, l'objectif étant de simplifier et d'optimiser nos procédures, tout en conservant le même niveau d'exigence en matière d'environnement. Par ailleurs, une démarche d'ensemble, à l'échelle des bassins de risque, est indispensable, et nous sommes aujourd'hui pleinement engagés pour accélérer avec pragmatisme la mise en oeuvre de la politique publique de prévention des risques d'inondation.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, je veux m'associer, en préambule, au nom de mes collègues du groupe socialiste et républicain, à l'hommage unanime rendu à nos militaires morts pour la France.

C'est donc qu'il y a un problème, monsieur le Premier ministre, que M. le Président de la République évacue d'un « revers de formule » : les Français seraient « pessimistes ». Mais comment pourrait-il en être autrement, quand ils considèrent que leurs difficultés sont mal comprises de leurs gouvernants, quand les solutions avancées reposent quasiment toujours sur la stigmatisation de telle ou telle catégorie :

Monsieur le Premier ministre, où est l'État, l'État protecteur, qui garantit la cohésion sociale, qui maintient le vivre-ensemble malgré les différences, qui apaise, qui rassemble son peuple, bref, celui qui redonnera l'optimisme, voire l'espoir, à nos concitoyens

Si je me suis engagé, sous l'autorité du Premier ministre, dans la mise en place d'un projet universel, c'est peut-être porté par le souffle de l'histoire, pour essayer de faire en sorte que le soutien de l'universalité

de la formidable exigence qu'avait exprimée Winston Churchill- la différence entre un politicien et un politique, c'est que, quand l'un s'occupe des prochaines générations, l'autre s'occupe de prochaines élections -, nous avons souhaité mettre en place nous avons souhaité mettre en place un système répondant à l'exigence d'équité- les mêmes règles pour tous -, faisant de la retraite le reflet du travail

! Je crois que, sur ce sujet, nous pourrions nous retrouver.

Ma question s'adresse au ministre de l'agriculture. Elle porte sur la crise sanitaire que traverse la forêt ; j'y associe notre collègue Anne-Catherine Loisier, présidente du groupe d'études Forêt Monsieur le ministre, la forêt traverse une crise sans précédent. Les conditions climatiques ont mis à mal les peuplements forestiers. On compte désormais près de 2,7 millions de mètres cubes touchés, toutes essences confondues ; les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté sont les plus frappées. En outre, depuis la sécheresse de 2018, la propagation du scolyte a explosé, entraînant un dépérissement massif. Les volumes d'épicéas scolytés

Le 8 octobre dernier, vous avez annoncé la mise en place d'un plan de soutien de 16 millions d'euros, pour valoriser le bois scolyté et replanter. C'est un début, mais, face à l'ampleur du désastre, cela s'avérera vite insuffisant. Comment ce plan se déclinera-t-il ? Cette tempête silencieuse qui frappe nos forêts françaises est aussi un véritable enjeu européen, puisque l'Allemagne et les pays d'Europe centrale sont eux aussi fortement touchés. À titre d'exemple, l'Allemagne vient de concevoir un plan de 800 millions d'euros sur trois ans. C'est donc une catastrophe économique, écologique et sanitaire. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire à court et à moyen terme ? La forêt a besoin d'une politique très ambitieuse : il est urgent d'évacuer le bois contaminé, afin de contenir la propagation, il est également nécessaire de réinvestir massivement dans nos forêts ; il y va de l'héritage que nous laisserons aux générations futures.

à la mémoire de nos soldats disparus tragiquement dans l'accident d'hélicoptère intervenu au Sahel, alors qu'ils étaient engagés en plein combat contre des groupes djihadistes armés. chers collègues, nos forces paient un lourd tribut à cette guerre qu'avec un courage et une abnégation sans limites elles livrent pour notre sécurité, celle des Français, mais aussi celle de toute l'Europe.

Avec une émotion toute particulière, nos pensées et notre affection vont ici à notre collègue, Jean-Marie, qui nous parlait si souvent de ce fils tant aimé, dont la vocation était le service de la France. Écoutons le message de son père, hier soir nous sommes dévastés, mais nous sommes fiers de lui » ; car, en vérité, ces treize soldats n'étaient pas là par hasard ; ils avaient choisi cet engagement au nom des valeurs, auxquelles ils croient, auxquelles ils croyaient. En cet instant, nous leur devons qu'il n'y ait pas de polémique. Nous leur devons respect, recueillement et reconnaissance. Ici, au Sénat, viendra sûrement le temps des interrogations. Elles sont légitimes. Peut-être aussi faudra-t-il un débat. Mais, aujourd'hui, aujourd'hui, nous savons que, face à une extension de la menace djihadiste vers les pays voisins, notre présence militaire est indispensable. Je dirai même qu'elle est incontournable, car, sans sécurité, inutile de croire au développement ou à plus de présence sur le terrain de l'État malien, déjà si défaillant.

sommets- sommet européen et sommet des nations occidentales de l'OTAN -, pensez-vous, monsieur le Premier ministre, pouvoir mobiliser plus encore nos alliés européens et occidentaux, afin qu'ils nous aident encore plus efficacement et qu'un tel drame ne se reproduise plus jamais- en d'autres termes, pour que Pierre-Emmanuel Bockel et ses compagnons d'infortune ne soient pas morts pour rien

je n'ai rien à ajouter à l'essentiel de l'intervention que vous venez de prononcer. Je mesure l'émotion de l'ami la parfaite compréhension que vous avez de l'ensemble de ces sujets, compte tenu des responsabilités que vous exercez au sein de la Haute Assemblée. Vous connaissez les militaires français, vous les voyez régulièrement, vous les auditionnez ici, vous les saluez, avec de nombreux sénateurs, sur les théâtres d'opérations

le sens de l'engagement profond et, en même temps, la très grande simplicité dans les rapports humains qui prévaut généralement lorsque l'on rencontre celles et ceux qui servent sous les drapeaux français. Bref, monsieur le président, comme beaucoup d'entre nous ici, vous les aimez.

vous l'avez dit, nous sommes au Mali pour d'excellentes raisons. Nous sommes au Mali pour garantir la sécurité de la France. Nous sommes au Mali pour accompagner des États partenaires et amis.

l'interroge. C'est ce que vous faites depuis longtemps et c'est ce que vous continuerez à faire. Il est légitime, normal, sain, dans une démocratie, qu'il en soit ainsi. Vous l'avez dit également, monsieur le président, nous devons faire en sorte que la France, qui n'est pas seule au Mali, puisse être plus accompagnée encore. faire en sorte que les mandats de l'ensemble des structures qui interviennent soient probablement mieux coordonnés. Nous devons faire en sorte que les objectifs politiques et opérationnels soient adaptés au fur et à mesure que la menace mute et se transforme. Il appartiendra au Président de la République de s'exprimer, après le temps du deuil, sur ce que nous pouvons faire pour convaincre nos alliés et nos amis européens que l'intérêt de l'Europe se joue aussi dans cette région. Il appartiendra à l'ensemble de la communauté nationale et des acteurs du débat public de convaincre nos partenaires sur place, les États du Sahel, qu'une partie décisive de la solution se trouve dans leurs mains

Union Centriste. Monsieur le ministre de l'agriculture, il ne vous aura pas échappé que, aujourd'hui, à Paris, comme dans un certain nombre de villes françaises, nos agriculteurs sont dans la rue. Après l'espoir suscité par la loi dite « Égalim » et les États généraux de l'alimentation, les agriculteurs de notre pays sont amenés à constater que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances qu'ils ont nourries et que, collectivement, nous voulons leur donner depuis tant d'années. Une réalité nous rattrape encore et toujours : celle des prix agricoles. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, elle relève de la responsabilité de votre Gouvernement

Pourtant, ce sont ces milliers de paysans qui nourrissent nos 68 millions de concitoyens, avec pour seul retour les attaques des doctrinaires environnementaux et animalistes Les agriculteurs font des efforts considérables. Ils ont acquis une grande capacité de remise en cause, comme peu de personnes dans notre société. Les pratiques agricoles évoluent pour améliorer la qualité des produits.

Malgré tous ces constats, le phénomène d'agri-bashing s'acharne, mitraille, harcèle l'agriculture de ce pays. Monsieur le ministre, comment redonner une raison de vivre aux agriculteurs ? Comment leur permettre de gagner leur vie ?

ont tout simplement marre du dénigrement permanent. Les agriculteurs en ont marre de se faire insulter lorsqu'ils épandent dans un champ. Les agriculteurs en ont marre des

nos agriculteurs sont aujourd'hui perdus, totalement perdus, et la colère qui s'exprime aujourd'hui à Paris et aux alentours est un cri. Monsieur le ministre, notre agriculture est en grande difficulté. Ma question est simple : comment comptez-vous répondre aujourd'hui à la détresse des agriculteurs descendus

je crois que la mobilisation d'aujourd'hui des agriculteurs- je vais devoir quitter le Sénat, parce que je les reçois tout à l'heure -va contribuer, avec le travail des parlementaires et du Gouvernement, à faire évoluer la situation.

Vous avez fait adopter la loi Égalim, censée sauver le revenu agricole, mais celle-ci ne porte que sur 20 % de ce revenu. La théorie du ruissellement ne fonctionne pas ! Vous dites soutenir la compétitivité des exploitations, mais la même loi augmente les charges. Le différentiel est devenu insoutenable, alors que nous n'avons jamais autant importé. Vous pariez sur la montée en gamme, mais vous soutenez les accords commerciaux qui ouvrent nos marchés à des produits ne répondant pas aux exigences de production. Je pense au CETA et à l'accord sur les viandes bovines américaines que le Parlement européen s'apprête à voter demain. Vous dites préparer l'avenir, mais vous laissez se préparer une PAC prévoyant une renationalisation des budgets, ce qui favorisera une concurrence intra-européenne mortifère. Monsieur le ministre, je crois sincèrement qu'il nous faut un grand projet de loi de programmation pluriannuelle agricole, qui nous permette parler de l'innovation, de la formation et des investissements durables, qui offrira un cap à nos agriculteurs et une ambition à notre pays et qui nous donnera confiance, à nous, Français, qui oublions trop souvent notre chance.

Que constatons-nous ? Malgré tous vos efforts de communication environnementale, le vernis se craquelle devant la suppression sans précédent du nombre d'emplois de fonctionnaires au sein de votre ministère. Rien que pour cette année, 2 500 postes disparaissent. Pour l'année 2020, ce sont 1 073 postes que vous supprimez ! Ce sont les fondements mêmes du service public de l'écologie qui sont mis en danger, jusque dans nos Pis, sur les trois années à venir, vous prévoyez de poursuivre cette destruction à la hache des effectifs, en supprimant près de 5 000 postes, soit 5 % des agents de votre ministère.

Vous embarquez le pays dans une politique publique paradoxale, où l'écologie est dans tous les discours, tout en sapant les moyens de l'État. S'il y a bien un secteur qui devrait être sanctuarisé, c'est bien celui de l'écologie Les collectivités territoriales, qui sont le fer de lance de la transition écologique, ont besoin du soutien de l'État pour l'ingénierie de projet, la logistique, la proximité. Combien de petits projets seront annulés parce qu'ils engageraient trop de frais de gestion ? Prenez garde de ne pas saborder les dynamiques vertueuses Les syndicats, toutes tendances confondues, vous ont pourtant alertée. Les membres du groupe socialiste et républicain souhaitent faire de même et vous demandent, à l'occasion du débat budgétaire qui s'ouvre cet après-midi au Sénat, de revoir votre copie, pour être à la hauteur d'une politique publique que les Français attendent de pied ferme.

le Président de la République et le Premier ministre l'ont clairement exprimé : l'écologie est l'une des priorités de l'acte II du quinquennat. Cette priorité suppose évidemment des moyens. C'est bien ce que traduit le projet de loi de finances pour 2020, avec une nette augmentation des crédits de mon ministère : plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour agir.

Je veille évidemment à ce que cet effort soit compatible avec la bonne mise en oeuvre de nos priorités. C'est pourquoi certaines missions, comme la biodiversité ou l'inspection des installations classées, sont préservées. Avant que nous en débattions tout à l'heure, je voudrais rappeler trois priorités portées par le budget de mon ministère.

autre grande priorité pour 2020 consiste en un effort sans précédent d'investissement pour les transports du quotidien, des transports plus propres, avec 3 milliards d'euros pour l'Afitf, ce qui est la traduction de la loi d'orientation des mobilités récemment adoptée. Enfin, nous allons accompagner notre politique en faveur de l'eau et de la biodiversité avec, notamment, la création de l'Office français de la biodiversité. Vous le voyez, la priorité est là et les moyens sont au rendez-vous

avec lesquels nous sommes en contact soutiennent le principe de l'universalité. Il est très clairement ancré dans l'esprit de tous que nous voulons bâtir un système où les mêmes règles s'appliquent à tous. Ils ont également parfaitement compris que, sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, nous voulions mettre en place un système équitable : à métier identique, retraite identique.

écologique et solidaire, le Président de la République s'est exprimé sur le dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques lors du congrès des maires. Vous en faites une interprétation tout à fait subjective, alors que le débat débute à l'Assemblée nationale. Nous ne souscrivons pas à votre proposition d'expérimentation sur les territoires volontaires, avec une mesure d'étape en 2023. Que de temps perdu ! Il y a urgence environnementale. Ne nous enlisons pas dans de faux débats. Le seul mot d'ordre qui tienne est de sortir du tout-plastique. Or le système de recyclage nécessite de toujours réinjecter de la matière première plastique dans la production. Je le dis sans ambages : vous ne prenez pas la bonne direction. Vous allez déséquilibrer un service public dont le modèle économique est en train de faire ses preuves, entravant, par voie de conséquence, l'action volontariste des territoires en matière environnementale. Vous participerez à toujours plus de plastique. Vous mettrez à contribution les consommateurs, qui vont payer plus et dégrader un peu plus l'environnement en se déplaçant aux points de collecte.

le projet de loi anti-gaspillage, porté par Brune Poirson et actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, est l'un des textes fondamentaux pour la transition écologique et solidaire que nous défendons. écologie du quotidien et transformation profonde de nos modèles de consommation. S'agissant du service public de gestion des déchets, qui est l'un des enjeux de ce texte, je voudrais réaffirmer très clairement et sans ambiguïté le rôle central des collectivités locales. Rien ne peut se faire sans elles sur ce sujet. Comme nous nous y étions engagés, nous avons de nouveau réuni, lundi dernier, les associations d'élus, en présence des organisations professionnelles et des ONG, pour évoquer le sujet de la consigne : nous nous sommes accordés sur une méthode pour atteindre l'objectif de 90 % de bouteilles plastiques collectées et recyclées dans dix ans. Cette méthode repose sur six engagements : la mise en place d'un groupe de contact entre l'État et les représentants des collectivités locales ; la définition d'une mesure objective des performances de collecte, de tri et de recyclage ; la garantie de mener à son terme l'extension des consignes de tri la réalisation, en 2023, d'un bilan pouvant conduire à la mise en place d'une consigne mixte pour recyclage et réemploi dans des conditions qui devront être précisées dans la loi

pour traduire ces engagements dans le projet de loi, à l'occasion de l'examen en séance publique, dans deux semaines, à l'Assemblée nationale. L'objectif est là. Nous avons, pour l'atteindre, une méthode partagée, dans laquelle la consigne jouera tout son rôle. remercie, madame la ministre, de votre réponse, mais, pour atteindre l'objectif, des solutions existent déjà dans les territoires qui ont mis en oeuvre la loi Grenelle. Il suffit que le Gouvernement fasse enfin respecter cette loi lors de l'examen du projet de loi Économie circulaire par notre assemblée, un excellent travail a été réalisé sous la houlette de Marta de Cidrac. Reconnaissez-le et soutenez-le

Les liens entre santé et nutrition sont de mieux en mieux connus, comme en témoignent aujourd'hui les recommandations nationales et internationales sur l'alimentation. Comme vous le savez, nous développons le Nutri-score, de façon à mieux alerter nos concitoyens et à les aider à être acteurs de la prévention en s'alimentant de la meilleure des façons possible. Nous savons que le risque de développer un grand nombre de maladies chroniques est lié à la manière dont nous nous alimentons. Je vous rejoins dans l'idée qu'il est important

Nous veillons à ce que l'information soit la meilleure possible, car nous disposons d'alertes sanitaires sur la qualité de ces produits, qui échappent à la réglementation.

jeudi dernier, vous avez lancé l'application numérique mobile « Mon compte formation ». Ce nouvel outil doit permettre à quelque 28 millions d'actifs de choisir, depuis leur smartphone, une formation pour obtenir des compétences supplémentaires, voire se reconvertir. Ce sont aussi 25 millions d'euros mis à la disposition des Français. J'ai testé cette application : effectivement, en moins de cinq minutes, munis du numéro de sécurité sociale, nous sommes informés du crédit en euros dont nous disposons pour financer une formation de notre choix, ainsi que des organismes agréés les plus proches, et ce sans demander d'autorisation spécifique ou remplir de longs formulaires. Si les Français s'en saisissent, une telle application pourrait permettre à la France d'investir dans ce qui fait le succès des pays aujourd'hui : les compétences. De surcroît, nos concitoyens auront la possibilité de s'épanouir en enrichissant leur parcours professionnel ou de réaliser enfin la formation rêvée. Cette démarche correspond à notre époque, où les citoyens veulent prendre leur avenir en main et ne plus se laisser dicter par d'autres la formation qui leur conviendrait le mieux. Avec cet outil, la formation devient, comme la santé, un droit fondamental. Le progrès technologique est plus que jamais- il faut vous en féliciter -un progrès social et économique. L'outil est là ; les Français doivent s'en servir. Aussi, madame la ministre,

cette transformation, j'ose dire cette révolution : la formation professionnelle. Depuis jeudi dernier, nous avons lancé, avec le Premier ministre, « Mon compte formation ». C'est un droit qui arrive directement à 25 millions de nos concitoyens. Aujourd'hui, ce sont les salariés et les demandeurs d'emploi ; en avril, ce seront aussi les 3 millions d'indépendants. Oui, c'est une révolution, car, aujourd'hui, il n'y a qu'un salarié sur trois dans les petites entreprises qui accède à la formation. Alors qu'un métier sur deux va se transformer dans les dix ans qui viennent, cet accès à la compétence, c'est la protection contre le chômage ; c'est la possibilité d'avoir une évolution de carrière, de changer de métier, de changer d'entreprise, de mener sa vie professionnelle. Oui, cette application répond à ces besoins en étant très simple, comme vous l'avez dit. En quelques clics, on peut découvrir ses droits, plus de 1 000 euros en moyenne. La moitié des Français disposent déjà de 1 400 euros. Ils auront 500 euros de plus chaque année, 800 euros s'ils ont un handicap ou s'ils n'ont pas de diplôme. On peut découvrir l'offre de formations : il y en a déjà plus de 140 000. Dans l'Hérault, votre département, 3 600 offres de formation sont déjà en ligne. Cela permet aussi, comme vous l'avez dit, de décider sans intermédiaire. C'est essentiel pour le futur. Comment le faire connaître ? D'abord, je voudrais dire que les Français ont répondu immédiatement très fortement. Il y a déjà eu 280 000 téléchargements à la Caisse des dépôts, qui est l'opérateur du ministère du travail dans les lancements d'applications de nouveaux services publics. C'est extrêmement élevé, et cela augmente d'heure en heure. Nous avons aussi prévu, avec Pôle emploi et Cap emploi, pour les demandeurs d'emploi, des conseils en évolution professionnelle gratuits, partout sur le territoire. Nous avons une campagne de médias, télévision et presse, qui démarre dimanche prochain.

plus de 30 000 sinistrés et plusieurs centaines de millions de dégâts. À la suite de ce drame, le conseil départemental, les intercommunalités et les communes des Alpes-Maritimes ont créé le Syndicat mixte inondations, aménagement et gestion de l'eau maralpin, dit Smiage, chargé de gérer le facteur inondation et de déterminer l'ensemble des travaux indispensables. En collaboration avec les services de l'État et les agences publiques, les aménagements urgents étaient donc parfaitement identifiés pour assurer la protection maximale des personnes et des biens. des pluies diluviennes inondaient de nouveau le Var et les Alpes-Maritimes, avec plus de 20 000 foyers sinistrés et d'innombrables effondrements et éboulements nécessitant des centaines de relogements. Pour beaucoup, il s'agit des mêmes victimes qu'en 2015.

et du logement (Dreal) freine, retarde et va jusqu'à bloquer la réalisation des travaux urgents et indispensables identifiés, sous prétexte de préserver des espèces dites protégées, batraciens ou plantes en tous genres. Et lorsqu'une étude se termine, elle en ordonne une nouvelle

aujourd'hui, qu'il est indispensable de créer une procédure d'urgence pour anticiper et faire face à ce genre de situations, qui se multiplient ? Par ailleurs, allez-vous donner des instructions à la Dreal pour faciliter les dossiers en cours et faire passer les vies humaines avant les espèces protégées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? aujourd'hui ? La parole est à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, vous l'avez rappelé, notre pays a été de nouveau durement touché par des intempéries le week-end dernier, avec onze départements en vigilance orange pour des risques divers de vents violents, d'inondations, de submersions marines. Effectivement, deux départements, dont les Alpes-Maritimes, ont été classés en vigilance rouge par Météo France. Je voudrais de nouveau exprimer toute ma solidarité aux familles et aux proches des victimes, et saluer la mobilisation exceptionnelle des forces de secours, des services de l'État, des collectivités et des opérateurs. s'est rendu sur place et il a pu constater cette mobilisation exceptionnelle. Face à ces événements, dont on sait qu'ils seront de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, il nous faut agir pour prévenir les conséquences des inondations. C'est ce que nous faisons avec les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI). C'est ce que nous faisons au travers des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI), avec des financements importants sur le fonds Barnier. C'est ce que font les communes

à mon ministère pour regarder ce qui peut aujourd'hui freiner la réalisation de ces programmes d'actions. Je disposerai très prochainement des propositions et je pense que nous aurons l'occasion d'en débattre. Il nous faut effectivement agir plus efficacement pour prévenir ces risques d'inondation, et c'est ce que nous allons faire.

après deux ans de réticences et de tergiversations, la convention de financement entre l'État et les collectivités locales pour la construction du canal Seine-Nord Europe a été signée par le Président de la République vendredi dernier. ce projet devient ferme et définitive, et l'État prend enfin sa part en s'engageant à apporter 1,1 milliard d'euros sur les 5 milliards d'euros du coût total. Si nous saluons cette formalisation, nous n'en demeurons pas moins circonspects. Sur la forme, d'abord. Certains parlementaires des Hauts-de-France n'ont pas été conviés et ont appris la nouvelle dans la presse. Bien qu'habitués au mépris du Gouvernement envers le Parlement, nous le déplorons fortement, la plupart d'entre nous ayant soutenu ce projet, souvent contre vents et marées. À ce propos, le Gouvernement est frappé d'amnésie lorsqu'il indique que ses prédécesseurs avaient « confondu les annonces et les actes ». Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire le canal n'existerait pas sans l'engagement du gouvernement précédent, qui a obtenu le financement à 40 % par l'Europe. Il n'existerait pas non plus sans l'acharnement, pendant plus de vingt ans, des élus et des collectivités territoriales, au premier rang desquels les élus socialistes. C'est votre gouvernement qui l'a suspendu en juillet 2017 Sur le fond, ensuite. Le Gouvernement a, en dernière minute et sans explication claire, fait adopter à l'Assemblée nationale un amendement au projet de loi de finances censé prévoir la part de financement de l'État.

Pouvez-vous aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, nous préciser les choses et nous certifier que cette augmentation sera exclusivement destinée à la construction du canal ? La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des transports. Monsieur le Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, vous avez rappelé que ce projet a beaucoup d'atouts. Il est vrai que c'est un projet qui est bon pour l'environnement, avec le transfert prévu de plusieurs milliers de poids lourds qui circulent actuellement sur l'A1. C'est un projet qui est bon pour l'économie portuaire et fluviale, non seulement pour la la région de Dunkerque, mais aussi pour les ports de l'axe Seine, que l'État s'emploie à renforcer depuis maintenant deux ans. C'est un projet qui est bon pour le territoire des Hauts-de-France, avec quatre plateformes multimodales qui vont être créées et connectées à cette nouvelle infrastructure, entraînant des emplois et de la croissance locale. Pour dire « oui » au canal, il fallait créer les conditions de crédibilité de ce projet. Vous l'avez dit, son coût a été réévalué à 5 milliards d'euros voilà deux ans, dans un exercice inédit de transparence et de sincérité budgétaire. Je peux vous affirmer ici que la sécurisation

Nous faisons confiance aux collectivités locales au travers de la société de projet qui sera régionalisée dès le 1 avril 2020, madame la sénatrice. Vous l'avez rappelé, l'Europe a été mobilisée à hauteur de 2 milliards d'euros sur ce projet. L'État veut par ailleurs que ce projet soit exemplaire

Enfin, et vous avez raison, madame la sénatrice, pour ce projet, il fallait une coalition d'acteurs et d'actions. À cet égard, je veux saluer les élus de tous bords, dont vous êtes, qui ont défendu avec opiniâtreté et détermination un projet que les Hauts-de-France attendaient depuis plus de quarante ans. Cependant, c'est notre gouvernement qui l'a rendu possible et donc irréversible, en signant la convention de financement, la semaine dernière, en présence du Président de la République, à Nesle. Cela permettra de donner les premiers coups de pioche vers Compiègne en octobre 2020 et de viser une mise en service à l'horizon de 2028. Nous en

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l'Assemblée nationale. Nous poursuivons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une augmentation des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables durables » de 9 % à périmètre courant, à un peu plus de 13 milliards d'euros. Il s'agit en fait d'une hausse en trompe-l'oeil des crédits de la mission, car trois mesures de périmètre gonflent artificiellement les crédits de la mission mission : les crédits dédiés au financement du bonus à l'achat d'un véhicule propre, inscrits jusqu'à présent sur un compte d'affectation spéciale, sont désormais inscrits sur le budget de la mission, pour près de 400 millions d'euros

dette de SNCF Réseau, pour 409 millions d'euros. Donc, madame la ministre, à périmètre constant, le budget de la mission s'élève en fait à un peu plus de 12 milliards d'euros, en baisse par rapport à l'an passé. Cette sorte de subterfuge du Gouvernement, qui vous permet de communiquer sur une hausse artificielle des crédits alloués à l'écologie, n'est, me semble-t-il, pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens s'agissant de l'urgence climatique.

Permettez-moi de douter que l'on puisse durablement agir sur davantage de missions avec moins de moyens financiers et moins de personnels pour conduire ces missions.

En réalité, 510 millions d'euros proviendront d'un redéploiement des interventions des agences de l'eau. C'est un joli tour de passe-passe que l'État opère. Je m'inquiète également de la

j'en veux pour preuve l'actualité récente de l'incendie de l'usine Lubrizol, qui nous rappelle l'importance des plans et des politiques de prévention. L'augmentation des risques liés au réchauffement climatique implique des besoins de financement croissants en matière de prévention. À cet instant, je veux rappeler que la question de la soutenabilité du fonds Barnier, lequel participe au financement de cette prévention, se posera dès 2020. la trésorerie du fonds va diminuer de moitié en raison du niveau élevé de dépenses et du plafonnement des recettes. Après ce constat d'ensemble, je vais vous présenter les enjeux auxquels font face certains opérateurs.

qui complètent les actions en matière de biodiversité qui seront conduites par les fédérations de chasseurs. Ce nouvel opérateur bénéficie d'un financement conforté pour assurer sa mise en oeuvre et d'emplois consolidés.

aux charges de service public de l'énergie, dont le montant est arrêté tous les ans par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), et qui représenteront près de 8 milliards d'euros

Madame la ministre, le Sénat a rétabli ce CAS, que les députés ont proposé de supprimer à compter du 1 janvier 2021, car il constitue un bon exemple de transparence, de suivi et de traçabilité concernant l'usage qui est fait du produit de la fiscalité écologique. Le programme « Énergie, climat et après-mines » porte, lui, plusieurs dépenses destinées à accompagner la transition énergétique des ménages. D'abord, le chèque énergie bénéficiera à près de 6 millions de ménages en situation de précarité énergétique en 2020.

390 millions d'euros sont également inscrits sur le programme 174 afin de financer une partie de la prime de rénovation énergétique à destination des ménages modestes en 2020,

car elle permettra d'assurer la contemporanéité du versement de l'aide avec la réalisation des travaux. Jusqu'à l'an passé, les aides à l'acquisition de véhicules propres étaient financées par le malus automobile, lequel venait alimenter un compte d'affectation spéciale.

La programmation financière de l'Afitf, annexée à ce projet de loi, prévoit 13,4 milliards d'euros sur la période 2018-2022 pour investir dans les infrastructures de transport, soit un peu moins de 2,7 milliards d'euros par an. C'est un effort financier très significatif de la part de l'État, puisque les crédits augmentent de 40 %. Pour 2020, les crédits de l'Afitf devraient augmenter de 502 millions d'euros, soit de 20,2 %. On aimerait y croire,

le budget n'ayant pas été de 2,6 milliards d'euros, comme annoncé, mais uniquement de 2,4 milliards d'euros, soit un écart de 204 millions d'euros, en raison de la baisse des recettes liées aux amendes de radar. Pour trouver les financements nécessaires, le PLF pour 2020 prévoyait, d'une part, de taxer le transport aérien en mettant en place une éco-contribution. Cette ressource n'est pas satisfaisante et nous avons souhaité l'amender en première partie. de diminuer de 2 euros par hectolitre le tarif réduit de TICPE des transporteurs routiers. Cette mesure, prévue à l'article 19, mettant en péril la compétitivité des transporteurs français, ...

Le Sénat est prêt à travailler avec le Gouvernement pour trouver des sources de recettes pérennes pour l'Afitf. Différentes pistes peuvent être envisagées. J'en citerai deux : affecter davantage de TICPE à l'Afitf, ce qui serait logique pour une taxe environnementale trouver un moyen de faire contribuer à l'entretien de nos routes les poids lourds étrangers qui ne font que traverser notre pays, sans même s'y ravitailler en carburant. Notre deuxième point d'inquiétude est le budget de SNCF Réseau.

Je ne reviendrai pas sur le mécanisme de reprise de la dette, qui ne pose pas de difficultés particulières. La solution retenue présente de nombreux avantages : elle ne change rien pour les créanciers de SNCF Réseau et ne se traduit pas par une dépense budgétaire de l'État, qui aurait creusé le déficit de 25 milliards d'euros. néanmoins veiller à ce que la dette ne se reconstitue pas. Or, si l'on en croit un journal du soir qui a eu connaissance de documents non communiqués à notre commission des finances,

Nous avons eu connaissance bien tardivement- le lundi de la semaine dernière -du rapport qui devait venir justifier les besoins de financement supplémentaire de la Société du Grand Paris En l'absence d'informations précises dans ce document, il ne nous est pas permis d'apprécier l'effet de levier des recettes supplémentaires qu'apporteraient ces deux nouvelles taxes. Par ailleurs, ce rapport laisse entendre que de nouvelles taxes devront être créées à l'horizon de 2024. Le plan de financement de la SGP doit être revu. On ne peut pas continuer à légiférer sur ce sujet au coup par coup. Concernant le programme 205, « Affaires maritimes », je ne reviendrai que sur un point : le financement de la SNSM, En 2020, la subvention octroyée par l'État à cette société atteindra 10,7 millions d'euros, un chiffre sans précédent. Cette hausse de 73 % de la dotation à la SNSM vise à accompagner l'association dans le renouvellement de sa flotte.

de transport conventionnés de voyageurs », compte tenu des efforts de réforme accomplis ces dernières années pour tenter de revoir en profondeur l'offre de trains Intercités et de lui donner un second souffle. La parole

sur les billets d'avion, nous pose beaucoup de questions. Nous estimons que cette taxe n'aura pas l'effet incitatif attendu, bien au contraire : c'est une taxe de rendement qui ne permettra pas de réduire les émissions de CO2 du secteur, mais risque d'avoir un effet de décroissance.

Nous savons aussi que la recherche aéronautique, l'incorporation de biocarburants et la conception d'avions électriques ou fonctionnant à l'hydrogène constituent des voies d'avenir. Je serais heureux que le Gouvernement nous éclaire sur la manière d'y parvenir. Nous savons bien que cela prendra du temps et que, bien évidemment, cette transition écologique ne se décrète pas,

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la loi Énergie-climat, qui est le fruit d'un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, vient d'être promulguée par le Président de la République.

Dans le même temps, la fiscalité énergétique croît de 4 milliards d'euros ; la part de la TICPE perçue par l'État augmente pour sa part de 11 %. La remise en cause d'incitations fiscales induit une charge pérenne de 1 milliard d'euros pour les professionnels. Dans ce contexte,

C'est par une fiscalité incitative, soucieuse de l'effort d'innovation des professionnels et du pouvoir d'achat des ménages, que nos modes de production et de consommation d'énergie pourront durablement évoluer.

qu'un effort fiscal et budgétaire suffisant nous permette d'atteindre l'objectif de neutralité carbone que nous avons voté, de manière supportable pour notre économie et pour les ménages.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cela fait plusieurs années que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

pour enrayer la dégradation du patrimoine existant et le remettre à niveau en une dizaine d'années. Au-delà du réseau géré par l'État, les travaux de notre commission ont montré que l'état des ouvrages d'art gérés par les collectivités territoriales était inquiétant et que ces collectivités ne disposaient, la plupart du temps, ni de l'ingénierie ni des moyens financiers suffisants pour les entretenir.

et d'intégrer dans les systèmes GPS des informations relatives aux ponts et à leur capacité, actualité malheureuse oblige ! Mais selon quel calendrier cela se fera-t-il, madame la ministre ? Un appui technique est nécessaire, mais insuffisant : les communes et les intercommunalités ne pourront pas procéder à l'entretien de leurs ponts sans aide financière. Madame la ministre, le Gouvernement est-il prêt à apporter une telle aide aux collectivités qui seraient dans l'obligation de remettre en état leurs ouvrages d'art en urgence ? S'agissant du dispositif de bonus-malus, nous regrettons que la hausse prévue du malus s'applique dans un contexte de restriction des aides à l'acquisition de véhicules propres, puisque les conditions d'octroi de la prime à la conversion ont été revues à la baisse cet été dans une logique budgétaire. Nous avons également entendu dire que le Gouvernement envisageait de diminuer de moitié le montant du bonus dont bénéficient les entreprises qui acquièrent un véhicule électrique, en le faisant passer de 6 000 euros nous confirmez-vous cette information ? Si elle était avérée, ce serait un véritable coup porté au renouvellement du parc automobile, étant donné que plus de 50 % des véhicules neufs sont acquis par des entreprises. Nous ne saurions donc l'accepter. Par ailleurs, je réitère mon opposition à ce que deux grilles de malus automobile soient appliquées l'année prochaine, comme le prévoit l'article 18, ce qui créera beaucoup de complexité, tant pour les professionnels que pour les consommateurs. Pourquoi demander aux membres de la Haute Assemblée d'approuver une grille de malus qui ne sera valide que trois mois ?

vois le canal Seine-Nord prendre forme et apporter un peu de tranquillité à cet axe autoroutier

sur les crédits relatifs aux transports ferroviaires, collectifs et fluviaux. J'ai toutefois pointé quelques sujets de vigilance, notamment en ce qui concerne la rénovation des petites lignes, dont on connaît l'état fortement dégradé, la diminution inquiétante du plafond d'emplois de Voies navigables de France, ou encore les moyens limités accordés à l'Autorité de régulation des transports au regard de l'extension de ses missions. Je souhaiterais d'abord vous faire part d'une remarque, madame la ministre, puis vous interroger sur le sujet du transport ferroviaire. D'abord, comme je l'ai annoncé, le budget de l'Afitf est en augmentation, de près de 500 millions d'euros, et nous ne pouvons que nous en réjouir : avec 2,98 milliards d'euros, ce budget se rapproche du scénario médian du Conseil d'orientation des infrastructures. Je tiens néanmoins à vous rappeler que l'année 2020 correspond à un pic pour l'Afitf et que, dès 2021, le budget alloué aux infrastructures de transports s'éloignera à nouveau des 3 milliards d'euros annuels prévus par le scénario 2 du COI. Lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités, notre commission avait regretté la trajectoire de dépenses retenue par le Gouvernement, sensiblement inférieure à celle du scénario 2 du COI, mais elle avait fait le choix

mobilités prévoit la définition d'une stratégie pour le fret d'ici au 1 janvier 2021, je souhaite vous interroger sur les mesures concrètes que vous comptez mettre en oeuvre rapidement dans le but de développer le fret ferroviaire.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis défavorable à l'adoption des crédits des programmes Elle a tout d'abord constaté que le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » poursuivra son assainissement financier, tout en maintenant un haut niveau d'investissements dans les programmes de modernisation des systèmes de gestion de la navigation aérienne. Par ailleurs, on ne peut que se satisfaire de l'augmentation de 20 % des crédits affectés aux lignes d'aménagement du territoire (LAT), ce qui permettra l'ouverture de nouvelles lignes, notamment entre Paris et Quimper. Comme l'a rappelé le récent rapport de notre collègue Josiane Costes, les LAT constituent des outils indispensables au désenclavement et à la cohésion des territoires ; elles doivent à ce titre être pérennisées. Ces motifs de satisfaction ne doivent pourtant pas masquer la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pavillon français, qui continue de perdre du terrain face aux compagnies étrangères, en particulier. Deux compagnies nationales, XL Airways et Aigle Azur, ont même fait faillite, occasionnant la suppression de près de 2 000 emplois directs. Le constat dressé au moment des assises du transport aérien, en 2018, n'a pas changé : les difficultés de nos compagnies s'expliquent en grande partie par leur déficit de compétitivité. À ce sujet, on ne peut que déplorer l'absence de cohérence de la politique du Gouvernement, qui avait allégé la fiscalité de l'aérien d'environ 120 millions d'euros dans dans la loi de finances pour 2019, avant de proposer dans le présent projet de loi de finances une hausse de la taxe de solidarité d'environ 180 millions d'euros afin de financer l'Afitf. Je salue à cet égard les amendements adoptés à l'article 20 du présent projet de loi de finances. Ces mesures permettront de compenser la hausse de cette taxe de solidarité par un allégement de la taxe de l'aviation civile et par un suramortissement sur l'impôt sur les sociétés pour les investissements de renouvellement des flottes. Je regrette cependant que la remise d'un rapport du Gouvernement portant sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France, prévue dans le projet de loi d'orientation des mobilités, ait été repoussée d'octobre 2019 à mars 2020. Le manque d'informations objectives en la matière affaiblit grandement la capacité du Parlement à débattre de manière éclairée sur le sujet crucial de la compétitivité du pavillon français. Pouvez-vous nous donner, madame la ministre, des indications quant au calendrier de publication de ce rapport très attendu ?

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la stabilisation, pour ne pas dire la stagnation, du budget des affaires maritimes et portuaires figurant dans le programme 205 et dans l'action n° 43 du programme 203, s'inscrit dans la continuité de la loi de finances pour 2019. Pour la deuxième année consécutive, l'État compensera à 100 % les dépenses de dragage des grands ports maritimes, ainsi que d'autres dépenses non commerciales de ces ports. L'administration des affaires maritimes poursuit sa modernisation avec l'acquisition de nouveaux équipements dédiés à la sécurité maritime. Plusieurs éléments positifs peuvent être relevés. Je pense à la subvention de 4,5 millions d'euros supplémentaires accordés à la SNSM. Si cette subvention ne résout pas l'enjeu majeur de la gouvernance de l'association, particulièrement relevé la mission commune d'information sur le sauvetage en mer, présidée par Corinne Féret, et dont le rapporteur était Didier Mandelli, elle constitue une aide bienvenue pour le financement des nombreux investissements auxquels doit procéder la SNSM pour renouveler la flotte de ses canots. Je pense aussi à la subvention exceptionnelle de 500 000 euros qui sera versée par l'État cette année pour soutenir la Fédération d'entraide polynésienne des sauveteurs en mer (FEPSM) pour l'acquisition d'un nouveau navire. Notre mobilisation sur ce sujet, au côté de notre collègue Lana Tetuanui, aura été déterminante ; je m'en félicite ! Le gouvernement polynésien apportera sa part, à hauteur de 500 000 euros, et la convention devra être signée rapidement pour que les travaux de construction du navire s'engagent dès le début de 2020. S'agissant des ports maritimes, le Premier ministre devrait présenter la nouvelle stratégie portuaire du Gouvernement à l'occasion du comité interministériel de la mer de décembre : il est temps Face au Brexit, face à la concurrence internationale dans le secteur portuaire, et face à l'avancée des « nouvelles routes de la soie » chinoises, il est plus que jamais nécessaire de bâtir une vision à moyen et long termes pour nos ports et leur infrastructure multimodale, et d'engager un plan d'action qui mobilise un ensemble d'instruments juridiques, économiques et d'investissement pour ancrer nos infrastructures portuaires dans les chaînes logistiques nationales et européennes et engager l'ensemble des acteurs dans une stratégie de conquête de parts de marché. D'ailleurs, je tiens à signaler à l'ensemble de mes collègues que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable met en place une mission d'information sur la gouvernance et la performance de nos ports. Madame la ministre, en 2019, notre commission avait émis un avis défavorable sur les crédits des affaires maritimes et portuaires, car le budget ne permettait pas de valoriser le deuxième territoire marin qui est le nôtre. Cette année, les manques sont, hélas, les mêmes. Toutefois, pour saluer les efforts réalisés dans l'urgence pour la SNSM et les sauveteurs de Polynésie française, mais également pour marquer une bienveillance à l'égard des futures annonces du Premier ministre sur la stratégie nationale portuaire, la commission, sur ma proposition, a souhaité émettre un avis d'abstention sur les crédits des affaires maritimes et portuaires pour 2020. Je conclurai mon intervention par une question : madame la ministre, quels moyens comptez-vous mobiliser pour construire une stratégie portuaire à la hauteur des enjeux économiques, numériques et de transition écologique, mais aussi de l'importance de notre zone

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme l'an passé, notre commission déplore l'absence d'effort budgétaire en faveur de la prévention des risques, ainsi que les baisses considérables d'effectifs imposées au ministère de la transition écologique et solidaire.

On ne peut donc que déplorer le maintien du plafonnement du fonds Barnier. Il faudrait au contraire revoir à la hausse les interventions de ce fonds, afin d'accroître l'effort de prévention face à l'amplification et à la multiplication des catastrophes naturelles, la prévention permettant de sauver des vies et de réduire sensiblement les besoins d'indemnisations.

En outre, le Gouvernement s'est fixé comme objectif une augmentation de 50 % du nombre de contrôles des ICPE d'ici à 2022. Selon les syndicats, sans augmentation des effectifs, c'est une gageure, sauf à réduire le temps consacré à chaque contrôle, y compris aux visites sur le terrain. Madame la ministre, comment entendez-vous atteindre cet objectif sans sacrifier la qualité des contrôles ?

Pouvez-vous nous préciser ce que cela implique pour le nouveau plan national santé-environnement ? Pour terminer, je relève que votre ministère est le deuxième le plus touché par les baisses d'effectifs, après celui de l'action et des comptes publics. Certes, chaque ministère doit contribuer à l'effort de maîtrise de la dépense publique, mais est-il cohérent, quelques mois après une déclaration de politique générale au cours de laquelle la réponse à l'urgence écologique a été présentée comme étant « le premier axe de la feuille de route » du Gouvernement, que le ministère responsable de sa mise en oeuvre continue de subir de telles suppressions d'emplois ? Vous l'aurez compris, mes chers collègues, au vu de ces observations, notre commission a émis un avis défavorable à l'adoption des crédits consacrés à la prévention des risques et à la conduite des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. La parole

le fait que la hausse des crédits de la mission soit en réalité due pour une grande partie à des mesures de périmètre ; deuxièmement, le fait que le ministère de la transition écologique et solidaire connaisse la deuxième plus forte baisse d'effectifs.

d'amélioration des prévisions et de prévention des catastrophes naturelles, seront-ils reconduits au-delà de 2022, afin que nous ne soyons pas très vite dépassés en matière de capacités de calcul notamment ? La prévision météorologique est essentielle, compte tenu

lequel deviendra à terme une prime plus simple et plus juste pour l'ensemble des Français ; le verdissement du parc automobile, grâce à la hausse de 50 % du bonus automobile ; la prime à la conversion ou encore le chèque énergie, doté de 822 millions d'euros en 2020, et le forfait mobilité durable.

Par ailleurs, ce projet de budget consacre la priorité accordée à la modernisation du réseau existant. Nous sommes nombreux, comme l'a rappelé notre collègue Didier Mandelli, à attendre la publication du rapport du préfet François Philizot sur les lignes ferroviaires de desserte fine des territoires. Ces petites lignes sont essentielles pour nos concitoyens, notamment dans les zones rurales et périphériques. Indispensables à l'aménagement d'un territoire donné, elles constituent une solution alternative à l'usage de la voiture. L'année 2020 marquera également la transformation profonde du groupe public SNCF, qui deviendra un ensemble de sociétés anonymes à capitaux publics. L'article 76 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit la première étape de reprise par l'État de la dette de SNCF Réseau, à hauteur de 25 milliards d'euros, en contrepartie d'efforts de productivité de la part de l'opérateur national. je salue le choix du Gouvernement d'une totale transparence sur le coût de cette reprise et de la création d'un programme budgétaire spécifique doté de crédits évaluatifs, le programme 355, « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État

J'en viens maintenant aux crédits du programme 205, « Affaires maritimes ». La France possède, vous le savez, le deuxième domaine public maritime au monde, ce qui constitue une véritable chance pour notre pays, car les enjeux sont considérables en termes stratégiques, géopolitiques, militaires, économiques, environnementaux et sécuritaires. De surcroît, la perspective du Brexit est source d'incertitudes. Le projet de budget que nous examinons finance les actions relatives à la politique de sécurité et de sûreté maritimes civiles, à la régulation sociale de l'emploi maritime, à l'action préventive en matière de sécurité maritime, au soutien à la qualité et au développement du pavillon français, ainsi qu'à la protection de l'environnement marin et littoral. Nous pouvons nous féliciter de la stabilité des crédits de paiement- ils s'élèveront à 157 millions d'euros pour 2020 -, tout comme de la hausse de 6,2 % du montant inscrit à la ligne budgétaire relative à l'action interministérielle de la mer, soit 13 millions d'euros.

Les hommes et les femmes de la SNSM sont de véritables héros du quotidien, et ils méritent toute notre reconnaissance. Tous sont très attachés à leur statut de bénévoles. Nous connaissons le courage et l'abnégation dont ils font preuve au quotidien. Une réflexion globale sur le modèle de la SNSM sera entreprise. Les défis sont nombreux : l'évolution des profils, la formation, l'entretien et le renouvellement de la flotte. La subvention publique en faveur de la SNSM passera cette année de 6 millions à 10,5 millions d'euros, comme le Gouvernement s'y est engagé. Il s'agit bien évidemment d'une excellente nouvelle, et je forme le voeu que ce financement soit pérenne. Le programme 113, « Paysages, eau et biodiversité », appréhende l'ensemble des actions liées à l'eau et à la biodiversité, qu'il s'agisse de la préservation des ressources et des milieux naturels terrestres et marins ou de l'aménagement concerté et de la protection des espaces, des sites et des paysages, en veillant au développement équilibré et durable des territoires.

Les risques naturels, les risques technologiques, les risques miniers et les risques pour la santé d'origine environnementale se concrétisent par des catastrophes aux conséquences humaines, économiques et environnementales majeures. Aussi convient-il d'assurer la transition de notre économie vers une économie circulaire et de réduire la vulnérabilité de notre territoire aux risques naturels, l'intensité des catastrophes étant accrue par le changement climatique. Le programme 181 porte également, depuis 2018, le financement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,

». La transition écologique et solidaire est un véritable projet de société, qui passe par une transformation de l'ensemble des secteurs économiques et par une mobilisation de tous les types d'acteurs : entreprises, collectivités, citoyens.

L'enfermement à Bercy nuit gravement à la lucidité ! La France ne peut pas conduire la transition énergétique sans ses opérateurs publics, en supprimant notamment des postes à l'Ademe. Elle ne peut pas préserver sa biodiversité en supprimant des postes dans les parcs naturels ou à l'Office français de la biodiversité

Globalement, les crédits de la mission augmentent de 1,1 milliard d'euros du fait de la transformation du CITE, du déploiement du chèque énergie et du début de la reprise de la dette de la SNCF. Nous ne nous en plaindrons pas. Nous nous félicitons même d'avoir inspiré le Gouvernement, sous la houlette de notre collègue Ronan Dantec, lors des débats budgétaires l'année dernière : l'instauration de l'écotaxe sur les billets d'avion permet enfin à l'Afitf de respirer un peu, son budget étant en augmentation de 11,4 %. Certes, Certes, nous continuons de demander que l'intégralité du produit de la TICPE serve à financer la transition écologique, et en premier chef les transports. Certes, nous souhaitons que le Gouvernement s'oriente vers le scénario 3 du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, lequel nécessiterait 4,5 milliards d'euros par an à l'horizon de 2023, mais nous saluons ce premier effort, qui appelle d'autres avancées, comme le retour d'une écotaxe en bonne et due forme. Il s'agit de faire participer le secteur routier aux financements des infrastructures afin de lutter contre la distorsion de concurrence entre la route et le rail.

nous nous désolons de ne toujours pas voir la couleur des 600 millions d'euros sur quatre ans promis pour la défense de la biodiversité. Si les crédits du programme 113 augmentent, c'est essentiellement pour compenser la baisse des recettes du permis de chasse, autre grande mesure en faveur de la biodiversité ... Au risque de me répéter, l'OFB n'a toujours pas les moyens de remplir ses missions.

Les visites ont, quant à elles, diminué de 40 %. Est-ce bien raisonnable ? Entre mesures de simplification, baisse des moyens financiers et pertes d'ingénierie publique, c'est toute l'évaluation et la démocratie environnementales qui sont mises à mal

a retenti sur tous les pavés du monde. De Paris à New York, en passant par Bangkok et Sydney, l'année 2019 aura été marquée par la volonté d'alerter et de dénoncer le manque d'action.

lutte contre la pollution de l'air, la prévention des risques climatiques, la protection de la biodiversité, la recherche et le développement d'énergies alternatives et efficientes, pour ne citer qu'eux. Le Gouvernement a fait, au cours des derniers mois, des propositions intéressantes. Je veux bien sûr parler de la loi relative à À cet égard, nous le savons tous, la question du financement, notamment des autorités compétentes en matière de mobilité, est centrale. Je souhaite toutefois saluer les efforts financiers proposés par l'État. Les crédits alloués aux infrastructures de transport

augmentation. Le changement climatique est l'une des principales causes des catastrophes naturelles, lesquelles vont devenir de plus en plus intenses. Nous allons donc devoir nous adapter et aménager durablement nos territoires. Des efforts supplémentaires devront être faits

je souhaite mettre en lumière le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Madame la ministre, nous devons rendre ce dispositif plus stable afin de gagner en efficacité et élargir son spectre. Il faut que l'État soit plus responsable et s'assure d'apporter des réponses dans des délais convenables. Le contrôle doit être accru pour éviter les dérives.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la première partie du projet de loi de finances pour 2020 a permis d'évoquer certaines mesures écologiques importantes, telles que la suppression progressive du tarif réduit de TICPE, la refonte des taxes sur les véhicules à moteur ou encore la suppression progressive du tarif réduit de TICPE pour les transporteurs routiers de marchandises. Que dire du volet dépenses concentré dans les crédits de la présente mission ? Deux orientations nous semblent particulièrement satisfaisantes. Premièrement, le projet de budget prévoit plusieurs mesures positives en faveur des transports ferroviaires, collectifs et fluviaux. La première d'entre elles, la sécurisation du budget de l'Afitf, était une mesure défendue par le Sénat lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités. Elle garantit la sincérité de la programmation financière des investissements de l'État dans les infrastructures de transport. L'augmentation des crédits relatifs à l'infrastructure ferroviaire traduit la mise en oeuvre des réformes récentes. Et la reprise de 25 milliards d'euros de la dette de SNCF Réseau par l'État permettra de mettre fin à la dérive de la trajectoire financière du gestionnaire d'infrastructure. L'effort d'investissement doit toutefois être poursuivi, compte tenu de la vétusté de nos infrastructures ferroviaires, et au regard de l'attention qui doit être portée à la préservation des dessertes fines du territoire. Deuxièmement, le budget traduit une stratégie équilibrée en ce qui concerne les transports aériens, associant l'assainissement du budget de la direction générale de l'aviation civile, une hausse des investissements et un accroissement du soutien aux lignes d'aménagement du territoire. Trois lignes de crédits nous semblent, en revanche, comporter des faiblesses préoccupantes. Tout d'abord, les moyens affectés à l'entretien du réseau routier et le soutien aux collectivités pour l'entretien des ponts sont insuffisants, ce qui est révélateur de l'état dramatique de sous-investissement de nos infrastructures. Par ailleurs, si l'objectif de « verdissement » de la présentation budgétaire doit être salué, les avancées concernant la biodiversité, la météorologie et la transition énergétique paraissent maigres. L'augmentation de 9 % des crédits de cette mission est davantage due à l'évolution du périmètre de ladite mission et à la compensation du manque à gagner de la réforme de la chasse pour le nouvel opérateur de la nature et de la biodiversité. à la diminution des effectifs du ministère chargé de l'environnement, elle semble en décalage avec la volonté du Gouvernement de faire de la réponse à l'urgence écologique le premier axe de sa feuille de route dans le cadre de l'acte II du quinquennat. Enfin, la stagnation des crédits consacrés aux transports maritimes semble peu compatible avec le développement d'une politique maritime ambitieuse, cela a été dit, en matière de compétitivité et de souveraineté, et alors que nous attendons la nouvelle stratégie portuaire que doit présenter prochainement le Premier ministre. l'heure où la Commission européenne fait de la relance de l'investissement sa principale priorité, et alors que la présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite mettre en place un européen, il est nécessaire d'accompagner le verdissement de notre budget par une évolution de nos règles de comptabilité

et de croissance, me semble appuyer une telle ambition. En conclusion, et sous réserve de ces remarques, le groupe Union Centriste votera les crédits de la mission « Écologie, développement et

En effet, chacun sait que les objectifs en matière de transition écologique et énergétique sont multiples, complexes, et tous plus ambitieux les uns que les autres. Je cite pêle-mêle : la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, la production d'énergies renouvelables fixée à 23 % en 2020, la neutralité carbone en 2050 ou encore la limitation à 1,5 degré de la hausse de température sur notre planète. Que de belles intentions ! Toutes sont censées nous conduire vers un monde meilleur ou plutôt, pour commencer, faire en sorte de préserver l'actuel

À ce titre, je suis pleinement en phase avec le rapporteur spécial Jean-François Husson, qui propose de ne pas adopter les crédits de la mission, notamment parce que la « fiscalité verte » présentée par le Gouvernement n'est en fait qu'une fiscalité de rendement déguisée visant à alimenter le budget général. Oserais-je rappeler que c'est en partie pour ce motif que le mouvement social a pris corps à l'automne dernier ? Avec mes collègues du groupe Les Républicains, je soutiens que la seule transition énergétique efficace est celle qui repose sur des actions très concrètes, progressives, financées et, bien entendu, consenties par la population. Sur ce point, je crains que ce budget ne soit un mauvais signal adressé aux Français. Ceux-ci ont besoin, et on les comprend, d'avoir la certitude que les taxes perçues contribuent effectivement à alimenter des incitations fiscales en faveur d'une transition. Las, le manque de simplicité et d'efficacité des mesures relatives à la fiscalité verte ne permet pas à l'ensemble de la population de consentir à modifier ses habitudes, à changer de véhicule ou à rénover son logement. Permettez-moi d'illustrer mon propos par trois exemples concrets. premier concerne la suppression du compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres », voulue par le Gouvernement, et celle du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique », votée à l'Assemblée nationale. Certes, il s'agit de mesures budgétaires un peu techniques, mais je suis convaincu que le message envoyé à l'ensemble des Français est extrêmement négatif ; les leçons de la crise que nous avons connue l'année dernière

La décision regrettable d'exclure les ménages des neuvième et dixième déciles aurait des conséquences immédiates, puisque ce sont eux, nous le savons, qui participent le plus à la rénovation du parc immobilier français.

après une année de mise en place, comme s'y est quasiment engagée Emmanuelle Wargon lors des discussions sur la première partie, à la suite de ma demande d'un rapport d'évaluation. Le troisième exemple porte sur la hausse du rendement de la TICPE- 1,4 milliard d'euros en 2020 -et le renforcement du malus automobile sans que le bonus soit augmenté dans les mêmes proportions. Nous avons, là encore, un beau cas de fiscalité non compensée, non accompagnée et non traçable pour l'automobiliste lambda. En séance, cette semaine, certains de nos collègues ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour imaginer des tas de nouvelles surtaxes sur les véhicules. Tout y passe, ou presque ! Le poids et- pourquoi pas ? -la taille ou le volume sont autant de pistes pour ceux qui ne comprennent pas que l'écologie punitive ne fonctionne pas et qui seraient mieux inspirés d'imaginer des incitations vraiment efficaces au sein de ce En matière de transition énergétique, nous attendons du Gouvernement qu'il fixe les priorités d'action pour le consommateur. Ce dernier conçoit que des efforts financiers, des changements de comportement et des travaux de rénovation seront sans doute sans doute nécessaires, mais il aspire également à une déclinaison pragmatique expurgée de toute empreinte idéologique. Malheureusement, l'exemple de ce projet de loi de finances et des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, parce que nous sommes confrontés à la menace de la plus grande catastrophe de tous les temps et parce que le compte à rebours a commencé, nous devons être autrement plus volontaristes que nous ne le sommes. Les rapports du GIEC ne sont-ils pas suffisamment alarmants ? L'idée est non pas de multiplier les discours anxiogènes, mais de parler vrai et d'agir juste,

Or je relève l'instabilité des aides, l'insuffisant accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, l'importance du reste à charge, des réticences des banques pour l'éco-prêt à taux zéro, l'insuffisante information des collectivités sur les dispositifs de la CDC. Force est de constater qu'il n'y a ni réelle dynamique ni dispositif innovant, si ce n'est des mesures à des échéances trop lointaines. L'urgence climatique attendra donc. Certes, la transformation du CITE en prime va dans le bon sens,

actuel, nous en saurons loin. Dois-je toutefois rappeler que nous sommes là sur le fondamental, tant pour le climat que pour l'environnement, la qualité de l'air et la lutte contre la précarité énergétique

crédits dédiés à qualité de l'air sont encore insuffisants, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France pour dépassement persistant des valeurs limites de dioxyde d'azote.

de la loi Climat-énergie, le véritable rendez-vous était celui du projet de loi de finances. Le Gouvernement avait l'occasion de présenter un budget plus volontariste pour opérer enfin le tournant attendu ; je regrette qu'il ne l'ait pas saisie. La parole

Le Président de la République lui-même n'est pas avare de phrases fortes sur la nécessité pour notre génération d'agir à la hauteur des enjeux face à l'Histoire. Nous aurions donc aimé, madame la ministre, retrouver le même élan, le même signal, dans le budget de l'écologie. Malheureusement, nous devrons encore attendre. D'après nos propres calculs, à périmètre constant, ce budget est en baisse de 214 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 20 millions d'euros en crédits de paiement. Les 800 millions d'euros supplémentaires annoncés sont liés principalement à la reprise par l'État de la dette de SNCF Réseau et à un jeu d'écriture sur le bonus-malus automobile. En d'autres termes, entre l'orthodoxie budgétaire, boussole de Bercy, et les grands enjeux environnementaux, où se joue la cohésion de nos sociétés dans les prochaines décennies, le Gouvernement a encore tranché, quitte à ce que cet esprit boutiquier de court terme ne joue au final contre le budget de l'État lui-même. Si on nous avait écoutés, par exemple, sur la nécessité d'un narratif différent sur l'augmentation de la contribution carbone-énergie, en jouant la répartition de cette recette dynamique entre les collectivités, les ménages modestes et l'État, votre budget s'en porterait bien mieux.

Les dépenses favorables à l'environnement, c'est, selon l'Inspection générale des finances, environ 35 milliards d'euros. Je crois que les Français ne comprennent plus et n'acceptent plus une telle situation. Ils sont prêts à l'effort, mais à la condition d'un contrat clair sur l'affectation des recettes. Je veux néanmoins me réjouir d'une décision : la réévaluation de la taxe sur les billets d'avion, dite taxe Chirac, en la rapprochant du prix du CO2 émis, comme nous l'avions déjà proposé dans un de nos amendements collectifs.

la ministre. Quand on s'attaque aujourd'hui à cette aberration que sont les SUV, nous retrouvons à peu près les mêmes arguments de défense d'intérêts économiques de court terme.

pour les opérateurs, la baisse est extrêmement importante. Elle touche très durement des établissements pourtant cruciaux pour l'adaptation au dérèglement climatique, comme Météo France, qui perd 95 équivalents temps plein, ou le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le Cerema, qui en perd 101. La même remarque vaut pour les inspecteurs des sites classés. Certes, leurs effectifs sont maintenus, mais seulement cette année, car la baisse a été importante les années précédentes. L'incendie de Lubrizol nous rappelle que l'État ne doit pas relâcher ses efforts en matière de contrôle. Les associations que nous avons auditionnées dans le cadre de la commission d'enquête avancent ainsi une baisse de 40 % des contrôles en douze ans. Nous proposerons donc un amendement visant à créer une trentaine de postes d'inspecteurs supplémentaires pour leur permettre d'y consacrer le temps nécessaire et augmenter ainsi les chances d'éviter de nouvelles catastrophes. Bien que la protection de la nature et de la biodiversité soit aujourd'hui une grande cause nationale, avec notamment l'organisation à Marseille- cela a été souligné -du congrès mondial de l'UICN au mois de juin 2020, le programme 113 ne répond pas à notre activisme international. les moyens qui permettent aux réserves naturelles d'assurer leurs missions de connaissances, de gestion et de surveillance de nos espaces naturels n'ont pas été réévalués depuis 2012. Les effectifs baissent, et ils sont en grande difficulté. Le plan Biodiversité a insufflé une dynamique d'extension de ces espaces, moyennant un engagement de créer à terme vingt réserves, dont une nouvelle cette année. Toutefois, les moyens humains ne suivent pas : on déshabille plutôt certaines réserves pour en permettre d'autres. Madame la ministre, je peux vraiment vous témoigner du désarroi sur le terrain des équipes professionnelles, qui considèrent ne plus avoir les moyens de leur action, pourtant centrale pour la biodiversité remarquable de notre pays. Je proposerai donc, là aussi, un amendement tendant à conforter leur capacité à répondre à cette mission tout à fait essentielle. Vous l'aurez compris, nous aurions préféré relever un tournant budgétaire décisif

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons plus douter de l'urgence de la transition énergétique à l'heure où se multiplient dans notre pays divers bouleversements résultant du changement climatique. Le groupe Union Centriste approuve le principe de la transformation du CITE en une prime : c'est une simplification bienvenue. De même, cibler cette aide en priorité vers les ménages les plus modestes constitue une mesure sociale qui mérite d'être saluée. Néanmoins, il reste regrettable d'exclure du périmètre du nouveau dispositif ceux qui réalisent 50 % des travaux de rénovation. Cela va à l'encontre d'une massification pourtant essentielle de la rénovation du bâtiment, secteur qui représente un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous déplorons aussi la réduction du périmètre des travaux éligibles au CITE. Pourquoi empêcher sa mobilisation pour les chaudières à gaz lorsqu'elles sont performantes ? Le gaz présente pourtant deux atouts de taille : cette énergie peut être propre et est produite en France. Il faut cependant noter les progrès obtenus durant les débats sur ces questions à l'Assemblée nationale. Je pense au geste consenti par le Gouvernement en rendant éligibles au CITE en 2020 les ménages des déciles de revenus neuf et dix pour les travaux d'isolation des parois opaques, mais également à la possibilité de mobiliser cette aide pour le premier achat d'un appareil de chauffage au bois performant ou encore pour les dépenses de rénovation globale pour les ménages des déciles de revenus un à

dont nous espérons la poursuite. Nous ne devons cependant pas nous en contenter. En effet, 20 % de ceux qui y ont droit n'y recourent pas, ce qui est encore trop. Eh oui ! Il convient donc de poursuivre les initiatives déjà engagées visant à faire connaître le dispositif. Une autre piste d'augmentation du nombre de sollicitations serait de permettre à nos concitoyens logés en Ehpad d'utiliser le chèque énergie.

Par ailleurs, nous saluons la volonté du Gouvernement d'accompagner la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et des centrales à charbon, matérialisant ainsi le respect des promesses du Président de la République. En revanche, je regrette que des moyens supplémentaires, notamment humains, ne soient pas attribués au médiateur national de l'énergie, alors que le nombre de litiges concernant la protection du consommateur ne cesse de croître : 17 000 en 2018 et déjà plus de 20 000 en 2019. J'en viens aux crédits du CAS « Transition énergétique ». Je note avec satisfaction le soutien accordé à la filière biogaz, qui doit continuer pour permettre à la France d'atteindre ses objectifs ambitieux de consommation d'électricité et de gaz issus d'énergies renouvelables. réforme du CAS « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale », votée lors de l'examen du projet de loi Énergie-climat, doit entrer en vigueur rapidement, pour permettre aux collectivités de s'adapter aux nouveaux défis posés par la transition énergétique, mais aussi pour que le critère de ruralité reflète mieux la réalité des territoires. L'examen des crédits relatifs à l'énergie Écologie, développement et mobilité durables » me conforte dans la conviction que le Gouvernement poursuit sur la voie de la transition énergétique avec détermination,

Grand. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs ». Ces mots étaient ceux du Président Chirac en 2002. On pourrait croire que les dix-sept années qui nous séparent de ce discours ont permis de prendre la mesure de l'urgence. Mais non ! La vérité est pire encore : notre maison brûle, et nous la regardons brûler ; nos digues cèdent sous la pression des éléments, et nous les regardons céder les abeilles meurent, et nous les regardons agoniser. Le monde tel que nous avons pu le connaître, celui dans lequel nous avons eu la chance de vivre quand nous étions enfants, est en péril. Nous vivons en plein ce que les scientifiques appellent la sixième extinction de masse. Si nous continuons à emprunter cette impasse, le pire est à envisager. Nous devons donc agir vite pour corriger cette trajectoire et espérer des jours meilleurs pour ceux qui nous succéderont. La France est une grande nation, fière de ses chercheurs.

tribune de la Haute Assemblée de trouver des moyens pour récompenser à la hauteur de leurs mérites nos scientifiques et éviter ainsi leur fuite vers des pays plus ambitieux dans le financement de la recherche. Le Président de la République semblait avoir pris la mesure des défis à venir lorsqu'il déclarait qu'il fallait rendre son lustre à notre planète. Deux ans plus tard, la France est-elle à l'origine d'une révolution écologique, elle qui sait si bien entraîner ses voisins dans son sillage et les inspirer lorsque sa trajectoire est bien définie ? Malheureusement, non ! Je ne suis pas partisane ; je suis objective, et je suis même désolée tel constat. Madame la ministre, les intentions du Gouvernement que vous représentez sont louables. Je vous crois honnête quand vous déclarez vouloir faire face à la crise écologique et environnementale qui nous guette. Alors pourquoi ne vous donnez-vous les moyens d'agir en fonction de vos ambitions ? Le Gouvernement proclame régulièrement que l'écologie est une de ses priorités. Les Français le réclament. En réalité, les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » diminuent de près de 230 millions d'euros cette année. Comment justifier cette baisse, alors que la plupart de nos concitoyens attendent des réponses ? Cet enjeu est indéniablement le plus important du XIX siècle ! En parcourant le budget que vous nous présentez, on remarque aussi une stagnation des moyens destinés à la prévention des risques. particulier au Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Comment accepter que ces moyens stagnent quand la métropole et l'outre-mer sont régulièrement en proie à des catastrophes climatiques ? En 2019, la France a connu des séismes, des inondations, des épisodes de neige exceptionnels, des tempêtes et des sécheresses hors du commun. Rien que ce week-end, les inondations dans le sud-est ont été effroyables, coûtant la vie à plusieurs de nos concitoyens. J'en profite pour réaffirmer que nous sommes de tout coeur avec les victimes. Perdre sa maison, son entreprise, ses biens ou, pis, la vie en raison de ces catastrophes climatiques, c'est terrible ces catastrophes naturelles et climatiques seront, à mesure que le temps passe, de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Les scientifiques sont unanimes sur le sujet. Il faut donc investir d'urgence

écologique de l'acte II du quinquennat. À première vue, cela pourrait relativement bien commencer, puisque le budget du ministère de l'écologie apparaît stable, grâce à l'astuce du compte d'affectation spéciale, ce qui a déjà été développé par mes collègues. Mais on déchante bien vite. Madame la ministre, comment comptez-vous respecter tous vos engagements et les faire appliquer concrètement avec une enveloppe à peu près constante et une nouvelle baisse importante d'effectifs au sein du ministère et de ses agences, comme vient de vous le demander mon collègue Joël Bigot lors des questions au Gouvernement ? C'est bien la survie de l'ingénierie publique dont il s'agit. Notre première inquiétude concerne le budget de l'Afitf. Nous ne pouvons que nous réjouir de le voir progresser dans le projet de loi initial, même si cela résulte de ce que je qualifierais de « bricolage estival » sur les 2 centimes de taxe sur le gazole des poids lourds faisant le plein en France et sur la taxe sur les billets d'avion.

La majorité sénatoriale vient une nouvelle fois de démontrer son refus de réparer une injustice fiscale entre les modes de transport pour assurer une transition écologique juste. Je pourrais également évoquer les paquebots de croisière polluants non fiscalisés. Notre deuxième inquiétude concerne Voies navigables de France. La hausse de son budget est bienvenue, mais la situation sociale résultant de la baisse des effectifs nous interroge. Nous ne pensons pas que l'effort budgétaire prenne en compte l'effet de la loi Didier, comme l'a révélé fort opportunément la mission d'information sénatoriale menée par Michel Dagbert et Patrick Chaize. Nous constatons d'ailleurs que leurs recommandations de qualité n'ont pas trouvé de débouchés dans ce projet de loi de finances. Je voudrais à présent aborder les routes. Outre l'insuffisance budgétaire pour éviter la dégradation de notre patrimoine, nous sommes toujours en attente de la publication du rapport Roche-Rapoport et de vos intentions relatives au réseau national. Surtout, madame la ministre, je tiens à vous faire part de notre très forte préoccupation concernant les financements destinés à notre système ferroviaire, tout particulièrement le budget de SNCF Réseau. Bien entendu, nous saluons la bonne inscription de la reprise de la dette de SNCF Réseau dans cet exercice budgétaire, mais où sont les fameux 10 millions d'euros d'investissements par jour promis par le Président de la République ? Car ce sont bien plus de 3 milliards d'euros qui sont nécessaires pour assurer la régénération du réseau dès 2020, il manquerait 250 millions d'euros pour respecter la dernière année de ce contrat de performance, selon une source syndicale, voire 345 millions d'euros, selon une autre source.

SNCF Réseau ? La problématique des « lignes modestes » n'est pas résolue. En deux ans, vous avez habilement réussi à éviter le débat, à tel point que certaines régions

a une vision comptable court-termiste. Mme la rapporteure spéciale semble faire sienne une telle méthode à propos des trains d'équilibre du territoire, puisqu'elle se satisfait du meilleur équilibre budgétaire sans faire état de la dégradation de l'offre ou de son transfert aux régions. À mi-mandat, nous pouvons dresser un constat : pour ce gouvernement, le ferroviaire n'est pas véritablement une solution. Des faits le montrent. Par ailleurs, je regrette le refus de la commission du développement durable d'accéder à notre demande d'audition des syndicats de cheminots en cette période particulière, puisque nous vivons un tournant majeur pour le modèle ferroviaire français avec l'application du nouveau pacte au 1 janvier 2020. Il n'y a jamais eu autant de démissions et de difficultés de recrutement dans ce secteur d'activité pourtant d'avenir pour la réussite de la transition écologique ! Cela est très bien illustré par une enquête interne la SNCF, commandée par la direction de l'entreprise elle-même. Elle fait apparaître que 63 % des salariés ne font plus confiance à leur entreprise pour améliorer leur avenir professionnel. Qu'en sera-t-il le 5 décembre prochain ? Pour pallier toutes ces difficultés, nous vous proposons de nouveau d'étudier l'idée de souscrire un grand emprunt, de généraliser le principe pollueur-payeur, de mettre à contribution les émissions carbone : des solutions jusque-là mais nous ne perdons pas espoir de vous convaincre afin de mettre chaque mode de transport dans son champ de pertinence économique et écologique. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons apporter des réponses aux problématiques de mobilités à deux vitesses. Madame la ministre, je suis au regret de constater que, malgré quelques progrès, ce budget est une nouvelle occasion manquée et ne répond pas à la double problématique de « fin du monde » et de « fin du mois ». Nous ne voterons pas les crédits de la mission.

Ce lundi, les circulations ferroviaires ont repris entre Béziers et Agde. Saluons l'engagement des agents de SNCF Réseau et des entreprises partenaires. Cette interruption de toute circulation durant un mois

arrêté en 1996, puis repris en 2007 avec des fonctionnalités différentes issues du débat public de 2009 ; quatre décisions ministérielles de 2010 à 2017 pour les études préalables devant mener à l'enquête publique avant d'être à nouveau stoppées en 2017. ans de tergiversations sur ce dossier ! La LOM, adoptée définitivement par l'Assemblée nationale, se base sur le scénario 2 du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Ce scénario prévoit une première phase de travaux sur le tronçon Montpellier-Béziers de 2028 à 2032 et une seconde entre Béziers et Perpignan de 2033 à 2037. Les événements climatiques à répétition sur le littoral méditerranéen nous obligent à reconnaître que ce calendrier n'est plus réaliste. En mars dernier, dans cet hémicycle, lors de l'examen de la LOM, je rappelais tout l'intérêt de ce projet structurant pour le développement de notre territoire. Il s'agit en effet du prolongement logique du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, qui vient de s'achever pour un coût de 1,8 milliard d'euros. Cette nouvelle ligne permettra de renforcer les mobilités du quotidien par un développement de l'offre de TER, mais également de répondre aux enjeux du développement durable par l'augmentation des capacités de fret. L'impact économique d'un tel chantier dans un département comme l'Hérault, rongé par le chômage, ne peut être négligé. Et l'Aude ! Cette ligne répond également aux enjeux européens d'interconnexion des lignes à grande vitesse françaises et espagnoles. que la ligne à grande vitesse Madrid-Barcelone-Figueras-Perpignan est déjà opérationnelle. Le dossier d'enquête publique est administrativement prêt : votre décision rapide, madame la ministre, de le lancer est unanimement attendue en Occitanie et marquerait un signal fort de la volonté de l'État d'avancer sur ce dossier. Annoncer un nouveau calendrier sans se préoccuper des financements serait mécaniquement irréaliste. La DUP en serait fragilisée. Avec le futur article 4 de la LOM, le Gouvernement est autorisé à légiférer par voie d'ordonnance dans un délai de deux ans- c'est très long ! -pour permettre la création d'établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre. C'est le cas du projet de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, dont le coût prévisionnel est de 5,5 milliards d'euros, dont 1,8 milliard d'euros pour le premier tronçon Montpellier-Béziers. La mise en oeuvre d'une société de financement permettra l'identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d'accélérer le le portage et la réalisation de cette grande infrastructure ferroviaire. Afin de perdre le moins de temps possible, pouvez-vous nous assurer d'un calendrier raisonnable pour la mise en place d'un groupe de travail sur la rédaction de cette ordonnance auquel la région Occitanie- sa présidente le répète souvent - souhaite activement participer ? participer ? Je ne résiste pas à l'envie de rappeler que l'État a su mobiliser en quelques jours plus de 10 milliards d'euros, que nous avons votés ici, pour satisfaire partiellement les « gilets jaunes », qui ne lui en sont pas pour autant reconnaissants. J'ai du mal à imaginer que l'État ne puisse tout aussi rapidement mobiliser les crédits nécessaires pour la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. La loi d'orientation des mobilités sera prochainement promulguée, mais les situations évoluent et les urgences s'imposent à nous. Dans ce domaine, il n'y a rien de plus vieux qu'une loi votée.

urgence que prend bien en compte le budget du ministère de la transition écologique et solidaire tel qu'il vous est proposé dans le projet de loi de finances pour 2020. En effet, après les amendements votés à l'Assemblée nationale, les moyens du ministère pour l'année 2020 s'élèvent à 32,202 milliards d'euros.

Ce budget s'inscrit bien dans la priorité donnée par le Président de la République à la transition écologique dans l'acte II du quinquennat. C'est une attente forte des Français, comme le grand débat national nous l'a montré. C'est aussi une nécessité et un défi. Le défi de la transition écologique pose finalement des questions simples dont les réponses peuvent être complexes : comment se loger, se nourrir, se déplacer ? Vers quels emplois s'orienter demain ?

domaine et de chacun de nos concitoyens. C'est pourquoi nos actions et nos moyens doivent accompagner ces derniers. C'est l'un des axes du budget que nous proposons, au travers du chèque énergie, de la rénovation énergétique des logements ou encore de la prime à la conversion. Une autre dimension fondamentale à prendre en compte est que la transition écologique n'est pas l'affaire d'un seul ministère. Elle constitue un objectif transversal pour tous les ministères, qui doit irriguer toutes nos politiques publiques. C'est ce que nous appelons le. Plus que le budget, ce le. Plus que le budget, ce sont les politiques mises en oeuvre par le Gouvernement dans le champ de la transition écologique et solidaire, et qui sont le reflet de nos priorités, que je voudrais présenter. Premièrement, l'eau et la biodiversité rassemblent 2,572 milliards

Nous allons créer le 1 janvier 2020 l'Office français de la biodiversité, qui permettra de simplifier notre organisation pour la préservation de la biodiversité et de renforcer l'efficacité des politiques publiques en coordonnant les actions et en développant ses partenariats territoriaux. Nous allons également créer un onzième parc national, le parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, dont la charte d'adhésion a été lancée il y a une dizaine de jours. Je le redis, j'ai souhaité que l'OFB soit préservé en 2020 de toute mesure de réduction de ses personnels. L'Assemblée nationale a accordé ETP supplémentaires, notamment pour la création de ce onzième parc. Grâce à la diversité des outils de classement et de protection, les aires protégées françaises couvrent aujourd'hui 29,5 % des terres et 22 % des eaux françaises. Le Président de la République a réaffirmé, à l'occasion du dernier conseil de défense écologique, l'objectif de 30 % pour les terres et les eaux, dont un tiers en protection forte.

Nous accueillerons à Marseille le congrès de l'UICN, qui traduira avant la COP15 Biodiversité en Chine, à l'automne, le positionnement moteur de la France à l'international, salué par tous nos partenaires. notre politique en faveur de l'énergie et du climat mobilisera 12,128 milliards d'euros en 2020. Nous poursuivrons le soutien aux énergies renouvelables financé dans le cadre du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique », notre premier poste de dépense avec 5,4 milliards d'euros. Avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous confirmons notre ambition de réduction de la consommation finale d'énergie, mais également le développement des énergies renouvelables avec des objectifs chiffrés. Depuis 2017, près de 3 000 projets ont été sélectionnés dans le cadre d'appels d'offres, dans le solaire, l'éolien terrestre, la biomasse, l'hydroélectricité et le fonds chaleur. Ces dispositifs ont permis la progression constante de la part des énergies renouvelables au sein de notre mix énergétique. Dans le mix électrique, la part des énergies renouvelables est ainsi passée de 19,6 % à 22,7 % entre 2016 et 2018. et 2018. L'Ademe, de son côté, sera dotée de près de 590 millions d'euros de crédits pour poursuivre ses appels à projets pour la transition énergétique et développer le fonds chaleur. La transition énergétique, c'est aussi aider nos concitoyens à franchir le pas d'un mode de vie écologique et plus économique. Le dispositif de chèque énergie, bénéficiant à plus de 5,8 millions de ménages, est largement adopté par les bénéficiaires potentiels : le taux de recours dépasse désormais les 80 %. En début de mandat, le Président de la République s'était engagé à retirer de la circulation 500 000 véhicules polluants grâce à la prime à la conversion. Cet objectif est d'ores et déjà rempli et même largement dépassé, avec presque 690 000 dossiers prévus à la fin de 2019, mais nous poursuivrons la mesure en 2020 : 405 millions d'euros y seront de nouveau consacrés, ainsi que 395 millions d'euros pour le bonus des véhicules électriques avec pour objectif désormais de retirer 1 million de véhicules polluants au cours du quinquennat. Comme nous nous y étions engagés, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui oblige aujourd'hui les ménages modestes à faire l'avance de trésorerie, sera transformé pour eux en prime directement touchée au moment des travaux. Grâce aux certificats d'économie d'énergie, les ménages peuvent être accompagnés, par exemple pour remplacer leur chaudière par un équipement plus performant en percevant une prime, qui peut aller jusqu'à 4 000 euros, et limiter le reste

un certain nombre de partenariats avec les premières régions. Quand j'entends dire que le Gouvernement baisserait le montant des aides à la rénovation thermique de l'habitat, je m'inscris en faux. En 2020, l'effort consacré à cette politique, essentielle pour l'efficacité énergétique, pour le confort, pour la qualité de vie et pour le budget des ménages, atteindra 3,5 milliards d'euros.

la politique de prévention des risques sera dotée de 532 millions d'euros. Ces crédits sont en très légère hausse par rapport à 2019. L'accident de Lubrizol rappelle que notre action dans ce domaine est une priorité. Une attention toute particulière est portée aux effectifs dédiés à ces missions. Les effectifs de contrôle des inspecteurs des installations classées seront maintenus l'an prochain, après avoir été en constante progression durant ces dernières années, et les effectifs de l'Autorité de sûreté nucléaire seront en hausse en 2020. La prévention des risques naturels majeurs est, de son côté, conduite en lien avec les collectivités. Le fonds Barnier, dont les montants d'intervention sont estimés à 180 millions d'euros en 2020, a été pleinement mobilisé lors des inondations dans l'Aude. Il accompagnera les collectivités et les ménages

présenté le 10 juillet 2019 en conseil des ministres, s'articule autour de quatre orientations que vous connaissez : stopper le gaspillage pour préserver nos ressources ; mobiliser les industriels pour transformer nos modes de production ; informer pour mieux consommer améliorer la collecte des déchets pour lutter contre les dépôts sauvages. Nos priorités budgétaires iront au renforcement des soutiens accordés par l'Ademe aux projets des collectivités pour valoriser leurs déchets et au contrôle des transferts transfrontaliers de déchets. les moyens alloués aux transports représentent 7,332 milliards d'euros. En forte hausse, le budget pour 2020 met en oeuvre les engagements pris dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Les audits sur les infrastructures que j'avais lancés en début de mandature nous ont donné une vision claire de leur état et des besoins pour améliorer la mobilité au quotidien de nos concitoyens. Nous nous sommes engagés dans la loi Mobilités sur une trajectoire financière pour l'Afitf : le budget pour 2020 y est conforme.

effort inédit en faveur de nos transports du quotidien est permis par le rehaussement de la contribution au financement des infrastructures du secteur du transport routier de marchandises et du secteur aérien, annoncé à l'issue du conseil de défense écologique du mois de juillet dernier.

est bien inscrite dans la programmation des infrastructures. Dès le vote de la loi, les réunions pourront commencer en vue de relancer la procédure de DUP. Comme vous l'avez souligné, la loi Mobilités offre la possibilité de créer des sociétés de projets pour accélérer les travaux si les collectivités le souhaitent. Pour nos concitoyens, nous avons l'objectif de tripler les déplacements à vélo d'ici à 2024. Pour y parvenir, nous engageons 350 millions d'euros sur sept ans dédiés au soutien des territoires. Nous avons également créé le « forfait mobilité » pour les salariés utilisant des modes alternatifs à la voiture. L'État le mettra en oeuvre pour tous ses agents dès 2020 pour un montant individuel de 200 euros. L'État confirme par ailleurs en 2020 son engagement auprès des ports, en sécurisant les moyens nécessaires à leur entretien, notamment en matière de dragages, et en poursuivant les plans de développement au travers des opérations inscrites dans les CPER. Enfin, la mission « Écologie, développement et mobilité durables » porte un nouveau programme destiné à financer la reprise de la dette de la SNCF. Cet engagement pris lors des négociations sur la réforme ferroviaire sera tenu. veux dire un mot sur les ouvrages d'art, sujet auquel, je le sais, la Haute Assemblée est particulièrement attentive. Pour le réseau routier national, je rappelle que l'effort global de régénération, était de 700 millions d'euros en 2017, sera de 850 millions d'euros en 2020. L'effort particulier sur les ouvrages d'art passera de 59 millions d'euros en 2017 à 79 millions d'euros en 2020 et atteindra 129 millions d'euros le budget consacré par mon ministère aux affaires maritimes s'élèvera à 296 millions d'euros. Je tiens à saluer particulièrement l'engagement des bénévoles et des personnels de la SNSM, qui, parfois au prix de leur vie, comme l'a tristement rappelé le naufrage au large des Sables-d'Olonne, apportent un concours indispensable à l'État pour la réalisation de secours en mer. Les subventions à la SNSM, qui avaient d'ores et déjà été doublées par rapport à la période précédente, sont désormais portées à 10,7 millions d'euros. Il s'agit

dont le rapport de M. Capo-Canellas avait montré l'importance, à hauteur de 18 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2019, soit 316 millions d'euros. Ces investissements sont notamment indispensables pour la fourniture de services performants et de qualité, en accord avec le nouveau plan de performance européen 2020-2024. En matière environnementale, le secteur est appelé à évoluer. Je rappelle que l'État consacre chaque année 135 millions d'euros à la recherche aéronautique civile, dont plus de la moitié au développement de carburants plus propres- les biocarburants -ainsi qu'au développement de motorisations électriques ou hybrides et hydrogènes à moyen terme.

mais aussi s'assurer que nos entreprises se positionnent sur les filières de la transition écologique. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce budget est à la hauteur pour mettre en oeuvre la priorité à la transition écologique et solidaire qui est celle du Gouvernement. Nous allons

programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables », afin de permettre à la Commission de régulation de l'énergie de signer un avenant visant à renouveler de façon anticipée le bail de l'immeuble qu'elle occupe rue Pasquier, à Paris. Quel est l'avis de

s'agit de compenser au bénéfice des collectivités, au travers des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ou des versements de TICPE, les charges résultant des transferts de compétences au titre de la gestion des fonds européens de développement rural transférés aux régions,

est à M. Roland Courteau. Comme le souligne, dans son rapport annuel de 2019, le médiateur national de l'énergie, près de 6 millions de personnes ont des difficultés à payer leurs factures d'électricité, de gaz ou de fioul et 7,4 millions de personnes vivent dans des « passoires énergétiques ». Toujours selon le médiateur national de l'énergie, en 2017, un tiers des ménages

pour la moyenne nationale. Le chèque énergie mis en place par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait notamment pour vocation d'aider les ménages à payer leurs factures d'énergie. Le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances pour 2019 d'augmenter la valeur du chèque énergie de 50 euros. Or la hausse des tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers en 2019 s'est traduite par une augmentation de 85 euros en moyenne pour les foyers se chauffant avec cette énergie, une somme particulièrement importante et pénalisante pour les ménages précaires, somme qui a annulé la revalorisation de 50 euros du chèque énergie. Force est de souligner que les populations fragiles sont les premières victimes de l'alourdissement des dépenses énergétiques contraintes, liées à l'augmentation des prix de l'énergie et de la fiscalité carbone. Pour ces raisons, nous souhaitons revaloriser le montant moyen du chèque énergie de 100 euros, afin que celui-ci permette aux ménages de vivre dignement sans renoncer par exemple à se chauffer. On peut estimer que le coût supplémentaire de cette augmentation est de l'ordre de 300 millions d'euros. Cela peut paraître élevé, mais nous avons de bonnes raisons de penser que les tarifs de l'énergie ne vont cesser d'augmenter, en raison de l'accroissement de la fiscalité écologique notamment. Il faut donc aider les ménages en situation de précarité, qui seront fortement impactés pendant la période de transition. Nous avons bien évidemment gagé notre amendement. Au regard des difficultés croissantes que rencontrent aujourd'hui les personnes en situation de précarité, le Gouvernement devrait lever le gage pour permettre une augmentation satisfaisante du montant du chèque énergie.

Il me semble important d'accompagner les ménages pour qu'ils puissent faire des économies sur leurs dépenses d'énergie. Ainsi, quand on change une chaudière à énergie fossile peu performante par un équipement à énergie renouvelable,

à M. Roland Courteau. Le projet de loi réforme, à son article 4, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, notamment en le transformant en prime perceptible dès le début des travaux de rénovation énergétique pour les ménages aux revenus modestes. Au total, 450 millions d'euros seront consacrés en 2020 au financement de cette nouvelle prime : 390 millions d'euros sont portés par le programme 174 et 60 millions

une ponction opérée sur un autre programme, mais nous sommes persuadés que Mme la ministre lèvera ce gage

Ce plan prévoit que des moyens dédiés à l'hydrogène seront mobilisés par l'Ademe pour permettre les premiers déploiements et que le Gouvernement mobilisera 100 millions d'euros à partir de l'année 2019. L'objectif du ministère de la transition et écologique et solidaire est d'atteindre un financement régulier de 100 millions d'euros par an en faveur de l'hydrogène, si les premiers déploiements sont concluants. L'Ademe a mené en 2019 deux appels d'offres en ce sens, mais les montants prévus à ce stade restent en deçà des 100 millions d'euros annoncés. Pour l'année 2020, le Gouvernement prévoit de proroger le soutien de l'Ademe au développement de l'hydrogène, sans plus de précision. Le bleu budgétaire relatif à la mission « Écologie, développement et mobilité durables » détaille le budget alloué pour 2020 à l'Ademe au sein de l'action n° 12 du programme 181. Avec un budget de 603 millions d'euros en 2019, le Gouvernement explique que ce financement permettra de démarrer les nouveaux fonds d'intervention- air, mobilité, hydrogène -et précise qu'en application du plan Climat, notamment pour accompagner les territoires dans la mise en oeuvre de leur plan de protection de l'atmosphère, l'Ademe poursuivra les programmes air et transport mobilités et sa dynamique sur l'hydrogène faible en carbone dans le cadre du plan Hydrogène. Cet amendement vise donc à doter

En juin dernier, dans un rapport d'information sur la sécurité des ponts, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a tiré la sonnette d'alarme sur l'état des ouvrages d'art du réseau routier français. J'associe bien entendu à mon propos le président de Si l'état des ponts gérés par les collectivités territoriales est particulièrement préoccupant, ce rapport rappelle également que les ponts gérés par l'État ont connu une dégradation lente, mais continue de leur état au cours des dernières années. À la suite de l'audit externe réalisé sur l'état du réseau routier national non concédé en 2018, le Gouvernement a lui-même indiqué que 7 % des ponts de l'État présentaient des dommages sérieux, avec, à terme, un risque d'effondrement. Nous le savons, après des années de sous-investissement, il est aujourd'hui impératif de mobiliser des moyens importants pour remettre en état ces ponts. En septembre 2017, un audit interne du ministère des transports a estimé à 110 millions d'euros par an les montants nécessaires pour améliorer l'état des ouvrages d'art de l'État et atteindre une situation normale d'ici à dix ans. Un constat similaire a été fait par le Conseil d'orientation des infrastructures, dans son rapport de janvier 2018. Quant au Cerema, il nous a indiqué que le budget consacré aux ouvrages d'art devait être porté à hauteur de 120 millions d'euros par an. Or le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d'y consacrer l'année prochaine 79 millions d'euros et la programmation des investissements prévue par la loi d'orientation des mobilités ne conduit à atteindre le montant de 120 millions d'euros qu'à partir de 2026. Le Gouvernement nous indique que cette trajectoire s'appuie sur le scénario 5 de l'audit externe du réseau routier, mais celui-ci ne permet, dans un premier temps, que d'enrayer la spirale de dégradation des ouvrages d'art, alors que l'enjeu est aussi de les remettre rapidement à niveau afin d'atteindre une situation satisfaisante. Par conséquent, cet amendement vise à augmenter de 40 millions d'euros les crédits dédiés à l'entretien des ouvrages d'art de l'État, pour les porter à 120 millions d'euros dès l'année prochaine, dans un contexte, évidemment, que l'on connaît tous.

Elle se verra ainsi confier le suivi de la création de nombreuses filières REP et la mise en oeuvre de la feuille de route pour l'économie circulaire. D'autres missions également, comme la mise en oeuvre du plan de déploiement de l'hydrogène, le nouveau fonds air-mobilité ou encore le service public de la performance énergétique de l'habitat nécessitent des moyens financiers adaptés.

Merci et à les rétablir à leur niveau de 2018. Le Cerema aide à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques du ministère de la transition écologique et solidaire. Il joue un rôle important dans le domaine des transports, des mobilités et de l'ingénierie, notamment en ce qui concerne les infrastructures comme les ponts, mais aussi de l'environnement. Parmi ses missions centrales figurent également la transition écologique et l'adaptation au changement climatique, des

les collectivités dans la mise en oeuvre de la compétence Gemapi. Or, depuis deux ans, cet opérateur a vu ses moyens chuter de près de 10 millions d'euros, soit 4,5 % de son budget total.

Au vu des missions importantes remplies par le Cerema, cette situation est anormale. En se basant sur le montant généralement admis de 50 000 euros par emploi, la baisse programmée de ces 101 ETP 101 ETP pourrait être compensée par 5 millions d'euros en 2020. Ce maintien des effectifs semble le minimum envisageable pour permettre à cet établissement de fonctionner normalement. L'amendement

Prévention des risques », à l'action n° 12, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, afin d'apporter une garantie au financement du plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique, présenté en juin 2018 par le ministère de la

Quelques semaines après l'événement survenu sur le site Lubrizol à Rouen, qui démontre la nécessité de maintenir les efforts en matière de contrôle et de prévention des risques, cette diminution de 6 millions d'euros est très mal venue. mal venue. Le dernier inventaire réalisé par le bureau d'analyse des risques et pollutions industriels (Barpi) du ministère de la transition écologique et solidaire, publié le 10 septembre dernier, a portant révélé que le nombre d'accidents industriels a augmenté de 34 % en deux ans, entre 2016 et 2018. Le rapport démontre que les accidents industriels causés par des événements météorologiques majeurs sont également en très rapide augmentation. Il apparaît dans le même temps que, en l'espace de dix ans, le nombre d'inspections a presque été divisé par deux. Dans ces conditions, la baisse des crédits dédiés à l'action n° 01 du programme 181

En effet, les conclusions des travaux du Barpi sont suffisamment alarmantes pour que des efforts financiers soient consentis en matière de prévention des risques. L'amendement n° Cet amendement de repli par rapport à l'amendement n° II-136 vise à limiter la baisse des crédits de l'Ademe en maintenant le montant de la subvention pour charges de service public à son niveau de l'année dernière, soit une hausse de 8 millions d'euros

de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse. Les modalités actuelles d'appréciation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation réhydratation des sols méconnaissent la gravité des phénomènes de cycles sur les sols argileux. Ce constat a d'ailleurs été établi par la mission d'information sénatoriale sur les risques climatiques. Les cycles de sécheresse et de réhydratation entraînent, à terme, la destruction des bâtiments édifiés de longue date sur ces sols.

Afin de parer aux conséquences les plus graves de ce phénomène, et en prévision d'une nécessaire réforme du système actuel de prévention et de réparation de ces dommages, cet amendement vise à créer un fonds d'indemnisation et de prévention des dommages liés à la réhydratation des sols argileux. Ce fonds, abondé dans un premier temps à hauteur de 3 millions d'euros, permettra de répondre aux premières urgences, de mettre en place des tours de table associant les acteurs territoriaux et les assureurs, de définir une stratégie de prévention de ces dommages et de faire évoluer les règles de droit commun de manière à mieux prendre en compte l'ensemble des sites.

dont l'importance ne cesse de croître à l'heure du changement climatique. Le rapport d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation de notre collègue Nicole Bonnefoy a mis en avant le rôle fondamental de cet opérateur de recherche et d'expertise dans l'anticipation et la gestion des aléas climatiques, mais aussi dans l'évaluation de l'impact du changement climatique. Pourtant, Météo France connaît une diminution drastique de ses effectifs depuis plusieurs années, et la tendance se poursuit en 2020, avec une diminution de 95 emplois. L'année dernière, l'opérateur enregistrait déjà une baisse de 62 emplois. La question de l'implantation de Météo France sur les territoires se pose donc nécessairement, particulièrement en zone de montagne ou en outre-mer. En effet, l'établissement devrait encore connaître la suppression de 475 emplois d'ici à 2022. Le présent amendement vise à maintenir le niveau de la subvention accordée à l'opérateur, soit une hausse de 1,7 million d'euros, ce qui pourrait correspondre au maintien de 34 emplois si nous estimons le coût moyen de ces derniers à 50 000 euros. Quel

est convaincu que l'hydrogène est un vecteur énergétique essentiel pour la transition écologique. C'est la raison pour laquelle, à la suite de l'annonce du plan Hydrogène, nous avons lancé trois appels à projets

Le premier appel à projets sur la mobilité a permis de retenir onze projets pour un montant de 50 millions d'euros ; les résultats des deux autres seront connus au début de l'année prochaine. Compte tenu de l'importance du sujet, nous avons d'ores et déjà décidé d'y consacrer de nouveau 50 millions d'euros en 2020.

S'agissant de la question des sols argileux et de l'impact sur les constructions, nous avons eu l'occasion d'échanger sur ce sujet lors du débat sur l'indemnisation des catastrophes naturelles.

Par ailleurs, en cas de sécheresse exceptionnelle, les dommages peuvent être indemnisés par le fonds « Catnat

qui vise à revenir sur la baisse de près de 6 millions d'euros des crédits alloués à la prévention des risques technologiques. Cette baisse semble motivée par le trop faible avancement des travaux réalisés dans le cadre des PPRT, les plans de prévention des risques technologiques. Beaucoup de ces PPRT sont désormais signés, mais, effectivement, il existe un problème

relatif à Météo France. De grands bouleversements sont devant nous. Les événements climatiques extrêmes sont en augmentation,

Cet amendement vise à maintenir le plafond d'emplois du ministère de la transition écologique et solidaire au niveau de celui de 2019. Nous considérons qu'il faut stopper la suppression d'emplois que connaît chaque année ce ministère. Il s'agit d'une impérieuse nécessité pour maintenir les compétences nécessaires à la mise en oeuvre de la transition écologique. Face à l'urgence climatique, ce ministère aura besoin de mobiliser de mobiliser toutes ses compétences et savoir-faire au bénéfice de la transition écologique. On ne peut plus continuer à s'enfermer dans une logique purement comptable, qui finit par compromettre l'avenir de notre planète. J'ajoute que la mise en oeuvre de la transition écologique nécessiterait au contraire le maintien de ces savoir-faire et la mobilisation de nouvelles compétences. Les suppressions d'emplois au sein du ministère se poursuivent chaque année, ce qui est particulièrement regrettable, d'autant

temps plein. Même si la transition écologique et solidaire est une priorité de l'acte II du quinquennat,

en préservant nos priorités- l'énergie, le climat, la prévention des risques et la biodiversité -et nous mettons davantage à contribution les fonctions support. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire que je ne pense pas souhaitable de baisser les crédits

aux préfectures et aux différentes directions départementales interministérielles. Cette décision entraîne en effet des transferts d'effectifs au profit de ces secrétariats généraux communs.

pour un responsable de programme. Au demeurant, la création d'un nouveau programme, qui serait l'un des plus petits du budget général, irait à l'encontre de l'objectif de simplification budgétaire. Pour autant, les dispositifs locaux d'accompagnement bénéficieront de 10,4 millions d'euros de crédits en 2020, alors que

Nadia Sollogoub. Par cet amendement, je souhaite donner aux agences de l'eau les moyens nécessaires pour honorer et solder leurs engagements auprès des particuliers qui se sont engagés dans une démarche de mise aux normes de leurs installations d'assainissement individuel sur la base de promesses d'aides financières.

Les élus communaux, dont je faisais partie à l'époque, avaient joué le jeu. La mission était ingrate et difficile : nous sommes allés chez nos administrés, nous avons fait de la pédagogie, nous avons promis des subventions, nous avons organisé des opérations coordonnées, nous avons fait réaliser des études préalables ... Maintenant

Il a été décidé, dans le cadre du onzième programme des agences de l'eau, de recentrer leurs interventions sur les actions les plus efficaces pour la reconquête de la qualité des milieux aquatiques et pour l'adaptation au changement climatique.

Il n'est pas dans mon tempérament de vouloir éviter les débats. J'ai eu l'occasion de dire que nous ne suivrions pas les préconisations du rapport Spinetta sur les petites lignes. L'État tient ses engagements dans le cadre des contrats de plan.